La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 5 avril a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

un rappel au règlement. Le Président de la République et son entourage ont laissé entendre que la France serait susceptible de s'associer aux États-Unis pour engager une agression armée contre le gouvernement de la Syrie. de la Syrie. Si cette agression se fait dans le cadre, légal du point de vue du droit international, de l'ONU, c'est quelque chose qui est tout à fait conforme, à ce qui se passe actuellement puisque l'engagement militaire de la France a été acté. En revanche, on a l'impression que M. Macron est prêt à bafouer le droit international et à passer outre aux décisions de l'ONU. Si tel était le cas, j'estime que la moindre des choses serait que le Parlement soit consulté pour que nous nous prononcions sur l'opportunité éventuelle de cette affaire. Pour ma part, je trouve que ce serait scandaleux. Au moment où nous recevons les pires des dictateurs, ceux d'Arabie Saoudite, l'un des pays arabes les plus arriérés,

conduite par M. Arūnas Gelūnas, président du groupe d'amitié Lituanie-France du Parlement lituanien. Elle est accompagnée par nos collègues M. Olivier Henno, président du groupe d'amitié France-Pays baltes, et M. André Reichardt, président délégué pour la Lituanie, ainsi que par M. Giedrius Mickūnas, ministre-conseiller de l'ambassade de Lituanie. La délégation vient d'être reçue par le groupe d'amitié France-Pays baltes et s'entretiendra cet après-midi avec notre collègue M. Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, et nos collègues membres du Bureau de la commission. L'année 2018 marque le centenaire du rétablissement de l'État lituanien, qui a été célébré au Sénat le 19 mars dernier, dans le cadre d'un colloque placé sous le haut patronage du Président du Sénat. Au nom du Sénat de la République française, je souhaite à nos collègues de Lituanie la plus cordiale bienvenue et forme le voeu que leur séjour en France contribue à renforcer encore davantage les liens qui unissent nos deux pays.

L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.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

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Polynésie française dispose de compétences étendues au titre de l'article 74 de la Constitution. Elle est dotée de l'autonomie. Dans un grand nombre de matières, c'est donc le Pays qui est chef de file. Il lui appartient de fixer des orientations et de définir les grands axes des politiques publiques. C'est à ce titre que la Polynésie française s'est dotée, par les lois du pays du 24 juin et du 23 février 2015, d'une réglementation des pratiques commerciales et d'un code de la concurrence. Cette initiative louable répond à des enjeux communs à tous les territoires d'outre-mer : faire vivre la concurrence est un défi dans des territoires insulaires- à l'exception de la Guyane, bien sûr -, souvent relativement coupés de leur environnement économique régional. Cette coupure peut être historique ; elle peut être aussi liée à la distance ; elle peut enfin résulter d'un niveau de développement sans commune mesure avec les territoires des environs. La Polynésie française a donc décidé de développer sa réglementation et des outils adaptés pour faire vivre cette concurrence indispensable à la lutte contre la vie chère. Car finalement, c'est bien le consommateur qu'il s'agit de protéger. À cette fin, la Polynésie a notamment institué une autorité polynésienne de la concurrence, l'APC, dotée d'un statut d'autorité administrative indépendante. Afin que cette autorité de la concurrence puisse exercer son activité, des dispositions complémentaires relevant de la compétence de l'État étaient nécessaires pour assurer l'effectivité des procédures de contrôle menées par elle. C'est l'objet de l'ordonnance du 9 février 2017, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, et entrée en vigueur le 30 juin 2017. Vous le savez, la Constitution prévoit une ratification expresse dans les dix-huit mois suivant la publication du texte, en l'occurrence avant le 10 août 2018. À défaut, l'ordonnance deviendra caduque. C'est l'enjeu du projet de loi soumis à votre examen. Sans revenir sur chacun des points de l'ordonnance en question, je crois utile de rappeler qu'elle permet notamment aux agents intervenant pour l'Autorité de procéder à des visites en tous lieux ou à la saisie de documents sur autorisation du juge des libertés et la détention du tribunal de première instance de Papeete. Elle permet aussi à ces agents d'accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et par les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française, sans se voir opposer le secret professionnel. Elle prévoit également les modalités de collaboration entre cette autorité locale et l'autorité nationale de la concurrence ou les services du ministère de l'économie : communication mutuelle des informations ou documents nécessaires, délégation de certaines enquêtes. L'APC disposera donc d'une panoplie d'outils de vérification et de contrôle identique à celle de l'autorité nationale de la concurrence. Les garanties en termes de voies de recours juridictionnel contre ses décisions seront également d'un niveau comparable. La commission des lois du Sénat a enrichi le texte par l'adoption de deux amendements. Le premier a étendu l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux membres des collèges et aux cadres dirigeants des autorités administratives indépendantes calédoniennes et polynésiennes. Cette mesure de mise en cohérence est la bienvenue. La commission des lois a également tenu à introduire dans le texte la détermination des délais de procédure et la fixation de la juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence. Ces éléments de nature réglementaire faisaient partie du projet de décret en Conseil d'État qui viendra compléter l'ordonnance, et dont la publication est prévue pour la fin du mois de mai. Je comprends toutefois que vous ayez voulu sécuriser le bon fonctionnement du dispositif institué. Mesdames, messieurs les sénateurs, avec ce projet de loi, l'État tente d'accompagner au mieux la Polynésie française dans l'exercice de ses compétences. Je vous remercie de l'attention que vous voulez bien lui accorder. La

En conséquence, sous peine de caducité, elle doit être ratifiée dans les dix-huit mois suivant sa publication, c'est-à-dire d'ici le mois d'août. Je veux d'abord rappeler le contexte de l'élaboration de cette ordonnance. En 2014, la Polynésie française a voulu se doter d'un droit de la concurrence moderne et cohérent, dans le cadre d'une économie insulaire de petite taille, dépendant d'un nombre limité d'acteurs économiques. Le marché polynésien ne représente en effet que 280 000 habitants, ce qui est propice aux monopoles ou, en tout cas, à une faible concurrence, au détriment des consommateurs. À cette fin, les autorités polynésiennes ont élaboré un code de la concurrence, directement inspiré du livre IV du code de commerce national, prévoyant notamment la création d'une autorité polynésienne de la concurrence, sur sur le modèle de l'autorité de la concurrence métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie avait déjà réalisé la même démarche peu de temps auparavant. D'une part, une loi du pays relative à la concurrence, votée en juin 2014 et promulguée en février 2015, a édicté les dispositions relevant de la compétence de la Polynésie. Ce texte a été entièrement validé par le Conseil d'État, qui en avait été saisi par une organisation professionnelle locale. D'autre part, une résolution de l'assemblée de la Polynésie française, adoptée en novembre 2014, a demandé à l'État de prendre les dispositions complémentaires relevant de sa compétence, en matière d'organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse. L'ordonnance que je vous invite aujourd'hui à ratifier est le résultat de cette démarche. Avant d'évoquer le contenu de l'ordonnance, je veux rapidement présenter l'autorité polynésienne de la concurrence, Les trois grandes missions de l'APC reprennent celles de l'autorité de la concurrence nationale : une fonction consultative, pour formuler des avis, soit d'initiative, soit à la demande des autorités locales une fonction de nature administrative d'autorisation des opérations de concentration économique, mais également- spécificité locale -des créations et extensions de surfaces commerciales une fonction de nature contentieuse de sanction des pratiques anticoncurrentielles, en particulier des cartels et ententes, mais également- autre spécificité locale -de certaines pratiques plus spécifiques à l'outre-mer, soit d'office sur proposition du rapporteur général de l'autorité, soit sur signalement d'une entreprise ou des autorités locales. Le président de l'autorité a été nommé en juillet 2015, les quatre autres membres du collège en septembre et le rapporteur général en décembre. Le 1 février 2016, le code de la concurrence de Polynésie est officiellement entré en vigueur et l'APC a rendu sa première décision en juillet 2016, sur un dossier de concentration dans le secteur hôtelier. L'autorité de la concurrence nationale a apporté un soutien particulier à la mise en place de l'autorité polynésienne. Le projet d'ordonnance n'a été transmis à l'assemblée de la Polynésie française qu'à la fin de l'année 2016 il a fallu deux ans pour répondre à la demande des autorités locales, pour rédiger une ordonnance de quatorze articles recopiant certains articles du code de commerce ... Même s'il n'a pas été rendu en temps utile, l'avis de l'assemblée était en tout cas favorable au projet. Publiée en février 2017, cette ordonnance appelait un décret d'application, qui devait être pris en principe avant le 30 juin 2017, madame la ministre, date butoir pour l'entrée en vigueur de l'ordonnance. À ce jour, plus d'un an après la publication de l'ordonnance, ce décret n'a toujours pas été publié Une telle carence est anormale, elle n'est pas respectueuse de nos compatriotes polynésiens. Que contient l'ordonnance ? Elle détermine les tribunaux compétents en Polynésie pour connaître des litiges en matière de pratiques anticoncurrentielles ; elle fixe les règles de prescription de l'action publique en la même elle précise les pouvoirs d'enquête des agents de l'APC, en particulier un pouvoir de visite et de saisie, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, et la possibilité de demander communication de tous les documents en possession d'une administration ou d'une juridiction elle fixe les voies de recours pour les décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles, devant le juge judiciaire, par dérogation aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Que ne contient pas l'ordonnance ? Les pouvoirs d'enquête ordinaires des agents de l'APC, ceux qui ne posent pas de problème de libertés publiques, car le Conseil d'État a considéré, lorsqu'il a examiné le projet d'ordonnance, que de telles dispositions relevaient de la compétence de la Polynésie. Or il y a moins d'un mois, le 14 mars 2018, l'assemblée de la Polynésie a adopté une nouvelle loi du pays pour modifier certains aspects du code de la concurrence, en particulier pour supprimer certaines prérogatives de l'APC en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et pour permettre au Président de la Polynésie d'évoquer les opérations de concentration afin de statuer lui-même si la décision de l'APC ne lui paraît pas satisfaisante. En revanche, curieusement, rien n'est prévu pour définir les pouvoirs d'enquête ordinaires des agents de l'APC ... Ce texte n'a pas encore été promulgué, compte tenu des délais de recours encore ouverts devant le Conseil d'État. Le vote de ce texte rend compte d'une certaine déception à l'égard de l'APC, voire d'une certaine contestation de décisions rendues en matière d'opérations de concentration sur un marché, encore une fois, très étroit, avec un nombre limité d'acteurs économiques. En tout cas, l'action de l'APC n'a pas conduit à ce jour à une baisse des prix, alors que c'était le premier objectif recherché. Néanmoins, du fait de la publication tardive de l'ordonnance, l'APC n'a pas encore pu rendre, à ce jour, de décisions sur des pratiques anticoncurrentielles. En tout état de cause, tout cela relève de la seule compétence des autorités polynésiennes. des autorités polynésiennes. Pour ce qui nous concerne, en tant que législateur national, il nous appartient simplement de ratifier l'ordonnance pour éviter sa caducité. La commission des lois y a apporté trois précisions : par analogie par analogie avec les règles déjà prévues par la loi pour l'autorité de la concurrence nationale, la commission a fixé les délais de recours contre les décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles et a retenu la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître de ces décisions

enfin, elle a rétabli l'obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie d'adresser une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, car cette obligation avait disparu en 2016, pour une simple raison rédactionnelle. Je vous propose donc, au nom de la commission des lois, d'adopter ce projet de loi de ratification ainsi modifié. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la Polynésie française fait souvent penser à de magnifiques paysages

! Ce qui est important pour la Polynésie française, ce territoire auquel nous sommes tous attachés, je crois, comme l'ensemble des Français et des Françaises y sont attachés,

Madame la ministre, madame la rapporteur, ce projet de loi y contribue assurément. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire- et c'était l'objet de l'ordonnance

celle du 25 juin 2014 et celle du 27 novembre 2014 -portant sur la concurrence ont été adoptées, mais leur objet était forcément limité puisque, comme vous l'avez dit, tout ce qui relève du code pénal ou du code de procédure pénale est encore aujourd'hui de la responsabilité de l'État. Il était donc très souhaitable que le droit de la concurrence puisse s'appliquer plus facilement, à travers des institutions adaptées. C'est l'objet de l'ordonnance qu'il nous est proposé de ratifier. Il s'agit de dire la compétence du tribunal de première instance de Papeete pour les litiges relevant des pratiques anticoncurrentielles ne concernant ni un commerçant ni un artisan de dire la compétence du tribunal mixte de commerce de Papeete pour les litiges concernant un commerçant ou un artisan ; de préciser les choses en matière de prescription et notamment de suspension de la prescription de l'action publique lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions compétentes ; il s'agit de préciser le pouvoir des agents de l'autorité polynésienne de la concurrence en matière de contrôle, notamment leur pouvoir d'enquête il s'agit de mettre au clair des dispositions spécifiques en matière de recherche d'identité, de telle manière que, lorsque les agents de l'autorité polynésienne de la concurrence ne pourront obtenir l'identité de la personne contrôlée, ils pourront en rendre compte à un officier de police judiciaire, qui pourra alors procéder à une vérification d'identité ; il s'agit de préciser les modalités et les garanties en matière de contrôles et de saisies par les agents de l'autorité polynésienne de la concurrence ; il s'agit, en outre, de préciser les modalités de recours devant la cour d'appel de Papeete, de préciser que le secret professionnel n'est pas opposable aux agents habilités de l'autorité polynésienne de la concurrence- bien entendu dans le cadre strict de leurs pouvoirs de contrôle de dire qu'il est nécessaire qu'un droit de communication des pièces du dossier d'instruction leur soit accordé enfin, des dispositions concernant le secret des affaires et la mise en oeuvre de la composition pénale viennent compléter ce dispositif. Mes chers collègues, je crois que nous nous retrouverons facilement autour de ces dispositions très techniques. Nous ne devons jamais oublier que nous les votons parce qu'elles sont nécessaires

madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, en 2014, la Polynésie française a voulu se doter d'un droit de la concurrence moderne et cohérent, dans le cadre d'une économie insulaire dépendant d'un nombre limité d'acteurs économiques. Le marché y est en effet très étroit et peu attractif, le territoire ne comptant que 280 000 habitants. C'est pourquoi la Polynésie française a élaboré un code de la concurrence, directement inspiré du livre IV du code de commerce national, lequel prévoit notamment la création d'une autorité polynésienne de la concurrence sur le modèle de l'autorité de la concurrence nationale. Une résolution de l'assemblée de la Polynésie française a demandé à l'État de prendre les dispositions complémentaires relevant de sa compétence en matière d'organisation judiciaire, de droit pénal, de procédure pénale et de procédure administrative contentieuse. Une loi du pays du 23 février 2015 a créé l'APC et édicté les dispositions de droit de la concurrence qui relèvent de la compétence de la Polynésie. Afin que cette autorité de la concurrence puisse exercer son activité, des dispositions complémentaires en matière d'organisation judiciaire et de procédure pénale sont indispensables. Ces mesures relèvent de la compétence de l'État et elles sont nécessaires pour assurer l'effectivité des procédures de contrôle. Tel est l'objet de l'ordonnance du 9 février 2017, entrée en vigueur le 30 juin 2017, qu'il nous est aujourd'hui proposé de ratifier. Les agents intervenant pour l'autorité pourront procéder à des visites en tous lieux et saisir tous documents sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete. Ces agents pourront accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et les services et établissements des collectivités publiques de la Polynésie française, sans se voir opposer le secret professionnel. Cette ordonnance exige un décret d'application, dont la rédaction a été finalisée et dont le Conseil d'État sera très prochainement saisi, pour une publication au début du mois de mai 2018. L'APC disposera alors d'une panoplie d'outils de vérification et de contrôle analogue à celle de l'Autorité de la concurrence au niveau national. Les garanties en termes de voie de recours juridictionnel contre ses décisions seront également d'un niveau identique à celui qui prévaut sur le plan national. La ratification de cette ordonnance est obligatoire dans un délai de dix-huit mois suivant sa publication, sous peine de caducité, en application de l'article 74-1 de la Constitution. Le délai expire en août 2018.

par analogie avec les règles relatives à l'Autorité de la concurrence nationale, pour ce qui concerne la fixation des délais de recours et la compétence de la cour d'appel de Paris. Cet amendement vise également à permettre la coopération entre l'APC, l'Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes- DGCCRF -, en matière d'enquêtes de concurrence sur leurs territoires respectifs. Le second amendement a pour objet de rétablir l'obligation, pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie, d'adresser une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe Les Indépendants voteront en faveur du projet de loi ainsi modifié par la commission des lois.

je ne serai pas long pour cette explication de vote, qui porte sur un sujet très spécifique, mais non moins important pour la Polynésie française. Lorsque l'on pense à la Polynésie, viennent d'abord à l'esprit des images de carte postale, la faune et la flore, la vanille, la perle de Tahiti, les écrits de Pierre Loti et les tableaux de Paul Gauguin. Voilà, en résumé, le mythe polynésien. Pourtant la Polynésie française se trouve dans une situation économique difficile. Avec la crise du secteur touristique, qui sévit depuis quelques années, les difficultés du secteur agricole, ou encore le faible développement de l'industrie, du fait de son isolement géographique, la Polynésie connaît un niveau de vie plus faible que la métropole. Le chômage, en particulier chez les jeunes, s'y est fortement accru au cours des dernières années. À ces problèmes s'ajoutent des caractéristiques plus structurelles, comme la part importante du secteur non marchand, une économie encore fortement administrée, avec le contrôle des prix, l'importation de la plupart des biens de consommation et un manque de concurrence entre les acteurs économiques.

l'huile de coco, ou coprah, et, surtout, les perles, qui trouvent leurs principaux débouchés en Asie, en premier lieu à Hong Kong, au Japon et à Singapour. Par ailleurs, la défiscalisation des investissements immobiliers est, comme dans les autres outre-mer,

en tant que collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution : son statut est spécialement régi par une loi organique datant de 2004, à l'instar du statut de la Nouvelle-Calédonie voisine- du moins vu d'ici L'assemblée de Polynésie peut ainsi voter des lois du pays, et l'archipel ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne, à la différence des départements et régions d'outre-mer. Toutefois, les dispositions prises à l'échelle nationale et concernant

Alors que nous discutons de ce projet de loi de ratification, les Polynésiens se préparent à élire, les 22 avril et 6 mai prochains, à l'assemblée de la Polynésie française pour les cinq prochaines années. L'examen de ce projet de loi de ratification de l'ordonnance du 9 février 2017 tendant à renforcer les pouvoirs de sanction en matière de concurrence survient donc en pleine campagne électorale.

L'organisation institutionnelle originale de cette collectivité d'outre-mer que constitue la Polynésie française en est l'un des exemples probants. En effet, depuis le renforcement, en 2004, du statut d'autonomie dont l'assemblée de la Polynésie française a la possibilité de voter des lois du pays dans le cadre de l'exercice de ses compétences. Ces actes, qui relèvent du domaine de la loi, sont soumis à un contrôle spécifique du Conseil d'État. C'est dans ce cadre que la Polynésie française s'est récemment munie d'une réglementation des pratiques commerciales et d'un code de la concurrence qui lui est propre, par des lois du pays du 25 juin 2014 et du 27 novembre 2014. Le caractère multi-insulaire de ce territoire, aussi vaste que l'Europe- faut-il le rappeler ? -, son éloignement des centres de production et la taille limitée de son marché favorisent de fait les oligopoles et les monopoles. Dès lors, les consommateurs se trouvent durement pénalisés. Comme son statut l'y autorise, la Polynésie française a également décidé de se doter d'une autorité administrative indépendante, l'autorité polynésienne de la concurrence, par une loi du pays du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1 février 2016. Toutefois, pour que cette autorité soit en mesure d'assurer pleinement sa mission et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs, il était nécessaire de compléter le dispositif par des prérogatives relevant de la compétence de l'État, particulièrement en matière de droit pénal, de procédure pénale ou de voies de recours. L'ordonnance du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française des dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, qu'il nous revient aujourd'hui de ratifier, s'y emploie. Les ajouts auxquels la commission des lois a procédé sur votre proposition, madame la rapporteur, chère Catherine Troendlé, vont dans le bon sens. Je pense notamment à l'obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes de transmettre des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 74-1 de la Constitution, cette ordonnance doit être ratifiée de façon expresse dans un délai de dix-huit mois, autrement autrement dit avant le 10 août prochain, sous peine de caducité. La procédure accélérée, engagée par le Gouvernement, ainsi que la procédure de législation en commission, d'une part, l'exercice du droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement en commission et, d'autre part, les explications de vote et le vote du texte en séance plénière, devraient nous permettre d'y parvenir dans les temps impartis. de ce projet de loi fait l'unanimité : permettre à l'autorité polynésienne de la concurrence, créée il y a tout juste deux ans, d'assurer pleinement sa mission, en complétant le droit local de la concurrence par des dispositions qui relèvent de la compétence de l'État.

ils permettront d'améliorer la lutte contre la vie chère, qui touche sévèrement nos compatriotes du Pacifique, tout comme ceux qui vivent dans les autres territoires ultramarins. C'est la raison pour laquelle les membres du groupe La République En Marche voteront en faveur

exprimer, nous ne disposons que de quelques minutes ... Le texte de cette ordonnance entend adapter à la Polynésie française les dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence. Si la loi polynésienne du 23 février 2015, entrée en vigueur le 1 février 2016, édictait un code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence calquée sur l'Autorité de la concurrence, il était nécessaire de la compléter pour les matières relevant de la compétence de l'État français. C'est l'objet de cette ordonnance, qui a été examinée selon la procédure de législation en commission. Je ne reviendrai pas en détail sur la position de mon groupe quant aux autorités administratives indépendantes, les AAI. Mais j'en dirai tout de même

a tendance à créer des situations de monopole ou d'oligopoles privés, d'ententes et de cartels qui pénalisent les consommatrices et consommateurs ultramarins. C'est pourquoi les membres du groupe CRCE sont favorables

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 23 février 2015, la Polynésie française édictait son propre code de la concurrence et instituait une autorité polynésienne de la concurrence : l'APC. Il s'agissait là d'une réforme économique d'ampleur, pour un territoire auparavant dépourvu de réel droit de la concurrence. En effet, ni les textes nationaux ni les règles du droit de la concurrence de l'Union européenne n'y étaient applicables, et seuls quelques textes épars réglementaient les pratiques et les relations commerciales. En 2015, la Polynésie française se dotait donc d'un droit de la concurrence moderne et cohérent, en créant une institution aux pouvoirs analogues à ceux de l'Autorité de la concurrence nationale, notamment quant au contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

C'est pour remédier à cette situation que l'ordonnance étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est aujourd'hui soumise à notre ratification. Composée de quatorze articles, cette ordonnance doit permettre à l'APC d'accomplir pleinement ses missions de contrôle et de sanction. Pour ce faire, elle complète les règles locales relatives à l'APC en matière de droit pénal, de procédure pénale, de procédure administrative contentieuse et d'organisation judiciaire. Les agents de l'APC disposeront désormais de pouvoirs d'enquête leur permettant d'effectuer des contrôles dans les locaux à usage professionnel. L'ordonnance attribue également à l'APC une compétence juridictionnelle pour les demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de pratiques anticoncurrentielles. Si elle fait siens ces différents objectifs, la commission a déploré la concomitance de l'examen du présent texte et de l'adoption, le mois dernier, par la Polynésie d'une loi qui modifie certains aspects du code de commerce et marque une certaine contestation de l'action de l'APC.

Cette loi du pays n'ayant pas encore été promulguée et étant encore susceptible d'être soumise au contrôle du Conseil d'État, il a été décidé de ne pas actualiser le contenu de la présente ordonnance.

dans un souci de sécurité juridique, la commission a prévu la compétence de la cour d'appel de Paris pour les recours à l'encontre des décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles tout en encadrant les délais de recours. Elle a également ouvert la possibilité d'une coopération en matière d'enquête entre l'APC et l'Autorité de la concurrence ou la DGCCRF. En permettant non seulement la transmission d'informations et de documents, mais aussi la conduite d'enquêtes, cette mesure devrait garantir un contrôle plus efficace des pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, elle mérite d'être saluée. Tout aussi louable est le rétablissement de l'obligation, pour les membres de l'APC et des autres autorités administratives indépendantes de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

règlement. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée s'apprête à débattre du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen,

Depuis la création des huit circonscriptions régionales en 2003, ce n'est pas la première fois que le rétablissement de la circonscription unique est débattu ici même. Vous le savez, une proposition de loi déposée par le groupe du RDSE a été adoptée le 23 juin 2010 par la Haute Assemblée pour rétablir cette circonscription unique. J'ai l'espoir que le Sénat adoptera une nouvelle fois un texte permettant de rétablir cette circonscription unique. En effet, si les options quant au mode de scrutin sont multiples, celle-ci m'apparaît comme la plus claire, la plus intelligible et la plus respectueuse du pluralisme politique. Elle est donc, à mes yeux, la meilleure pour nos concitoyens. Je sais, bien sûr, que tous ici n'approuvent pas cette vision. Mais, je le sais aussi, c'est dans un état d'esprit constructif que nous abordons tous ce débat.

: vous savez que, dès l'élaboration de ce texte, le Président de la République et le Premier ministre ont veillé à consulter l'ensemble des formations politiques dans le cadre d'une démarche de coconstruction législative. Mesdames, messieurs les sénateurs, si le Gouvernement a retenu l'option de la circonscription unique, ce n'est donc pas du fait du hasard : c'est bien parce que la majorité des groupes politiques avaient, avec lui, un diagnostic commun. commun. Au-delà des différences de sensibilités et de positionnements que les formations politiques peuvent présenter au sujet de l'Union européenne, je crois que nous sommes tous d'accord pour affirmer que la situation actuelle

Que l'on soit pour plus ou moins d'Europe, que l'on soit pour une Europe fédérale ou pour une Europe des nations, que l'on soit pour davantage d'intégration ou pour de nouveaux élargissements, l'on ne peut se satisfaire de si faibles taux de participation, qui minent la légitimité des députés européens et, finalement, affaiblissent la démocratie. Il est évident que le mode de scrutin n'est pas l'unique cause de la hausse de l'abstention- il faut le reconnaître.

-de dialoguer avec nos concitoyens sur le terrain pour comprendre que le découpage en huit circonscriptions, sans cohérence historique, politique ou administrative, a contribué à brouiller le débat entre enjeux européens, enjeux nationaux et enjeux locaux. Il fallait donc agir pour inverser cette tendance, et ce dans un délai court puisque, par tradition républicaine, le mode de scrutin n'est pas modifié dans les douze mois précédant une élection. C'est ce que le Gouvernement entreprend avec ce projet de loi.

Si le Gouvernement ne l'a pas retenue, ce n'est pas, comme on a pu l'entendre parfois, pour des raisons politiciennes, mais parce que le débat aurait certainement été perturbé par des enjeux étrangers à la nécessaire confrontation des idées et des projets relatifs à l'Europe.

de raisons juridiques, et notamment de risques constitutionnels. Non, madame ! La création d'une circonscription ultramarine aurait pour effet de garantir aux seuls électeurs ultramarins de disposer d'une représentation sur une base territoriale, tandis que le reste des électeurs ne bénéficieraient pas d'une telle spécificité. En résulterait un risque d'atteinte au principe d'égalité devant le suffrage. Au-delà des risques juridiques, la création d'une circonscription spécifique à l'outre-mer pose question sur le plan des principes. Une telle option ne manquerait pas d'être légitimement contestée par d'autres régions. Au reste, certains représentants français au Parlement européen, élus en 2014 dans la circonscription d'outre-mer, ne sont eux-mêmes pas favorables à la création d'une circonscription ultramarine, ... Lesquels ? ... qui marquerait une différence avec le reste de la Nation et qui affaiblirait l'intelligibilité du scrutin pour les électeurs. Dès lors, la meilleure option- nous en sommes convaincus -était bien la circonscription nationale unique.

d'abord, cette solution est soutenue par la majorité des partis politiques. Or, vous le savez, nous voulons toujours rassembler le plus largement possible face aux grands choix stratégiques qui engagent le pays.

c'est ce qui a principalement emporté notre décision -, nous sommes convaincus que ce mode de scrutin permettra d'intéresser davantage nos concitoyens à des élections qui sont de plus en plus décisives pour leur destin individuel comme pour leur destin collectif.

et la réalité des territoires. En tant qu'élue locale, vous connaissez mon attachement à ces sujets. Mais, si j'ai soutenu en 2010 la proposition de loi du groupe du RDSE, c'est, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que je suis, comme citoyenne de l'Europe, depuis longtemps convaincue que la circonscription unique est la meilleure solution. Pourquoi ? Parce qu'elle permettra de proposer aux Français des débats clairs, avec des options nettes sur la confrontation des projets européens.

inscrites dans le présent texte. Nous en débattrons lors de l'examen des différents articles. Pour l'heure, je souhaite évoquer plus particulièrement les modalités de répartition du temps d'antenne lors de la campagne officielle pour les élections européennes, lesquelles ont suscité de nombreux débats. lors des discussions à l'Assemblée nationale : il était de la responsabilité du Gouvernement de modifier le dispositif existant pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 31 mai dernier. Si nous n'avions pas modifié le dispositif, nous aurions laissé perdurer un système producteur d'injustices et nous aurions pris le risque d'une nouvelle censure. censure. Bien sûr, nous nous y refusons. C'est pourquoi nous avons élaboré ce dispositif équilibré reposant sur un triple mode de répartition, dont la dernière fraction corrective sera mise en oeuvre par le

Il existe donc un risque réel de vide juridique si nous ne prenons pas rapidement les mesures législatives adéquates. C'est pourquoi le Gouvernement a fait le choix d'emprunter ce vecteur législatif pour soumettre au Parlement un dispositif alternatif dont les principes sont identiques à ceux qui ont prévalu pour élaborer le dispositif de la campagne officielle des élections européennes. Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà de ce projet de loi, le Président de la République et le Gouvernement portent, vous le savez, des ambitions fortes pour l'Europe. Ces ambitions, le Président de la République les a exprimées lors de son discours de la Sorbonne, le 26 septembre dernier. Elles visent notamment à faire émerger un véritable espace public européen ce qui implique notamment qu'un débat politique émerge également à l'échelle européenne. Les négociations menées actuellement pour permettre la création d'une circonscription européenne unique et des listes transnationales s'inscrivent pleinement dans ce cadre et se poursuivent. Vous le savez, à l'occasion d'un vote le 7 février dernier, le Parlement européen n'a pas retenu le principe des listes transnationales pour les prochaines élections européennes, malgré un vote favorable en commission. Le Gouvernement a pris acte de ce vote, mais reste néanmoins très engagé pour faire aboutir ce projet, qui a déjà reçu le soutien de plusieurs de nos partenaires. Dans la perspective des élections européennes de 2024 et indépendamment du prochain scrutin, il continuera à défendre cette idée, car elle est la seule à pouvoir renforcer la démocratie européenne. Dans ce même état d'esprit, le Gouvernement entend poursuivre le combat pour refonder l'Europe et la rendre plus démocratique. C'est tout le sens des consultations citoyennes qui seront lancées dans quelques jours dans toute l'Europe. En France, l'ensemble du Gouvernement, mais surtout les acteurs de la société civile, le monde associatif, les entreprises, les partenaires sociaux, les collectivités y participeront, afin d'entendre les préoccupations, les attentes, les espoirs,

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous connaissez tous la fameuse phrase de Jean Monnet : « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Par ce texte, par les actions que met en oeuvre ce gouvernement, c'est bien ce but que nous visons : unir les Français, d'abord, autour de la belle idée européenne, autour de représentants qui porteront haut la voix de la France au Parlement de Strasbourg

qui fait que la voix de notre continent est écoutée et respectée partout dans le monde. La parole

président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat est convié à examiner une nouvelle fois le mode d'élection des parlementaires européens français,

les attitudes critiquables de certains parlementaires européens, qui ne se pliaient pas à un travail intensif de représentation et de communication avec le terrain et la population, il m'a semblé légitime de dire que le contraire existait aussi,

européens et énonce trois principes essentiels. Le premier est un système de listes à l'intérieur de chaque nation, laissant le choix entre des listes nationales complètes ou des listes réparties par circonscription.

Par ailleurs, notre tradition électorale, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé à plusieurs reprises, est de laisser la plus grande liberté dans la composition des listes et de ne pas contraindre les organisations politiques à structurer leurs listes selon un mode obligatoire.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, ce texte est l'occasion de nous demander quelle Europe politique nous souhaitons. Depuis sa création, sans interruption, ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'objet politique non identifié a posé une question de légitimité aux États et aux peuples. Je crois profondément que cet enjeu de légitimité est l'une des sources des maux de l'Union européenne et qu'il ne pourra y avoir d'avancées ou de réformes européennes sans que cette question centrale soit tranchée. Nous avons essayé beaucoup de choses pour que, enfin, le processus de construction européenne devienne légitime aux yeux des citoyens, qui avaient placé leur foi et leurs attentes dans l'État-nation Beaucoup d'entre nous ont tenté de rendre l'Union européenne plus démocratique, plus transparente, plus efficace. Force est de constater que, si nous n'avons pas totalement échoué, nous n'avons pas réussi non plus. Nos petites touches impressionnistes, nos petits pas- chers à Jean Monnet -visant à rendre l'Union européenne plus légitime n'ont pas été compris des peuples, qui n'y ont souvent vu que barbouillage ou petits arrangements. L'affaire Selmayr, que j'ai dénoncée devant la Haute Assemblée, participe de ce triste paysage que l'Union européenne s'offre parfois à elle-même. Un symptôme mesurable de ce désenchantement persistant se trouve dans la participation en chute libre aux élections au Parlement européen, Alors que les pouvoirs de ce dernier n'ont fait que se renforcer au fil des ans, la participation aux élections européennes a reculé de 46,8 % en 1999 à 42 % en 2014. Le Parlement européen est devenu ce qu'Hannah Arendt appelait « un pouvoir sans autorité », c'est-à-dire, en démocratie, un pouvoir privé de légitimité aux yeux des citoyens. La question que nous nous posons est donc la suivante : la mise en place de circonscriptions régionales en 2003 a-t-elle permis d'enrayer ce phénomène d'éloignement démocratique, a-t-elle permis de rapprocher les citoyens européens de leurs représentants ? Force est de constater que, depuis 2003, trois élections ont passé et que rien n'a changé. Le sentiment de non-représentation persiste chez nos concitoyens. Or ce panorama démocratique morose n'est pas une fatalité. Après tout, le slogan de la campagne des premières élections au Parlement européen au suffrage universel, en 1979, était déjà : « L'Europe, c'est l'espoir. Aujourd'hui, il nous faut retrouver cet espoir, provoquer un véritable choc démocratique pour l'Union européenne, afin de créer ce que Jürgen Habermas appelle un « espace public européen Le texte que nous examinons constitue un pas modeste dans cette voie, mais il contribuera, à mon sens, à rendre le débat européen plus présent et plus visible aux yeux des Français il permettra de mettre les grands dossiers de la politique européenne au premier plan des discussions ; il forcera chacune des forces politiques de ce pays à se positionner clairement, ce qui n'est pas encore gagné il permettra de donner de la lisibilité à un mode de scrutin assez opaque et méconnu par nos concitoyens ; il permettra, enfin, de porter au Parlement européen des députés plus forts et plus responsables face à leurs homologues européens, qui sont, pour la plupart, déjà élus sur des listes nationales.

alors que la politique nationale et la politique européenne ne sont pas des sphères séparées, comme on veut souvent nous en convaincre, mais constituent les deux faces de la médaille de l'intérêt général. Tout cela est positif. Nous soutiendrons par conséquent ce texte en l'état, mais cela ne suffira pas à réenchanter le projet européen. Il faut aller plus loin sur le chemin d'une véritable légitimité européenne. Tout d'abord, il faut trouver les moyens de faire en sorte que la composition de la Commission résulte d'un choix démocratique et non de petits arrangements entre États.

être mieux contrôlées. De même, l'opacité des manoeuvres entre États ne doit pas être remplacée par des arrangements entre les partis. Enfin, selon moi, le dernier pilier de la légitimité européenne doit être la proximité. L'éloignement des institutions et des parlementaires européens est une des causes du désenchantement des peuples. Paradoxalement, il me semble que l'ancien système de circonscriptions interrégionales, en raison de sa complexité et de son manque de lisibilité, n'a pas contribué à instaurer cette proximité. Le retour à la circonscription nationale doit aller dans ce sens, avec une représentativité plus forte des candidats et des engagements plus contraignants pour les parlementaires. La bataille de la légitimité, mes chers collègues, est la mère de toutes les batailles en Europe. Nous ne la gagnerons qu'en faisant preuve de courage politique et en acceptant, une fois pour toutes, qu'une Union européenne plus puissante et plus intégrée offre la promesse d'une France plus forte et plus influente. La parole

des États-nations au profit d'un magma européen. Ceux qui, comme moi, pensent que l'Europe supranationale, c'est l'Europe de la chienlit, ne peuvent pas soutenir cette proposition.

désaccord : la répartition du temps de parole. Il est scandaleux que, dans une démocratie, des candidats à une élection ne disposent pas des mêmes moyens et soient traités de manière discriminatoire.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les dernières élections législatives italiennes et, plus récemment encore, le scrutin qui s'est déroulé le week-end dernier en Hongrie sont des indicateurs effroyables du déclin de l'enthousiasme européen à travers le continent. Ici et là, les partis eurosceptiques gagnent du terrain et menacent l'équilibre pacifique qui se construit en Europe depuis plus d'un demi-siècle. C'est dans ce contexte inquiétant que le Gouvernement nous propose de préparer le prochain renouvellement du Parlement européen, selon une philosophie qui ne nous est pas étrangère. Vous vous en souvenez, dès 2010, sur l'initiative du groupe du Rassemblement Social et Démocratique Européen, la Haute Assemblée avait voté le rétablissement de la circonscription unique, mesure ne disparaisse dans les limbes de la navette parlementaire. Il a fallu huit ans pour que cette idée ressorte des cartons et que nos collègues députés l'adoptent des deux mains. Mieux vaut tard que jamais Vous ne serez donc pas étonnés d'apprendre que nous restons convaincus de la nécessité de cette réforme. Depuis le traité de Lisbonne, les règles françaises de désignation des membres du Parlement européen ne sont plus adaptées aux nouvelles prérogatives de ces parlementaires. Comment expliquer que des élus, dont le rôle est dorénavant déterminant, soient si mal identifiés par nos concitoyens, que leurs travaux fassent l'objet d'une si faible médiatisation et ne préoccupent que quelques spécialistes ?

À titre personnel, j'ai été convaincue par les débats qui se sont déroulés en commission des lois : la protection des intérêts des territoires d'outre-mer revient, comme celle des intérêts de tous les territoires de l'Union européenne, à l'ensemble des membres du Parlement européen. S'ils le désirent, les citoyens résidant dans ces territoires pourront orienter leurs votes vers les listes qui feront de l'outre-mer une priorité. Plusieurs de mes collègues soutiendront, au contraire, la création d'une circonscription spécifique pour l'outre-mer, conformément à la liberté de vote qui régit notre groupe. Plusieurs d'entre nous auraient souhaité que la possibilité de recourir à des listes transnationales figure dans le texte, nonobstant la portée peu normative de cette disposition. La réforme de l'acte électoral européen est toujours en discussion et cette évolution nous paraît nécessaire pour renforcer la démocratie européenne et faire émerger des groupements politiques transnationaux, susceptibles de défendre des projets politiques pour l'ensemble des citoyens européens. Nous soutenons tous les efforts du Président de la République en ce sens. Cette évolution n'est pas incompatible avec l'attachement à la République qui est le nôtre ni avec le rétablissement d'une circonscription unique qui nous est aujourd'hui proposé. Elle est au contraire en totale cohérence avec notre défense de la démocratie parlementaire. rapprocher l'Union européenne du citoyen en renforçant la légitimité du Parlement européen. Si nous nous apprêtons à voter ce texte, nous regrettons toutefois que son examen se fasse dans le cadre de la procédure accélérée, qui ne nous permet pas d'avoir des débats plus longs sur les moyens à développer pour sensibiliser pour sensibiliser davantage nos concitoyens aux enjeux européens. De plus longues réflexions auraient, par exemple, permis de se pencher sur une meilleure conciliation du principe d'égalité devant le suffrage et de l'objectif d'intelligibilité des débats lors de la campagne européenne. Si l'on peut comprendre la volonté du Gouvernement de limiter le temps de parole minimal attribué à chaque liste de candidats quand de telles listes se multiplient, l'établissement d'un système de parrainage aurait pu constituer une solution alternative, plus respectueuse du pluralisme auquel nous sommes très attachés. La question de l'éducation des jeunes générations d'Européens est également occultée. Elle est pourtant cruciale. Lors des dernières élections européennes, 73 % des électeurs français de moins de trente-cinq ans se sont abstenus. Depuis sa création, l'école républicaine a toujours eu pour ambition de former nos jeunes, de leur permettre non seulement d'exercer un métier, mais également d'exercer convenablement leur citoyenneté. C'est pourquoi nous présenterons un amendement visant à renforcer la dimension européenne de l'enseignement moral et civique, en particulier au collège. D'autres réflexions pourraient également être conduites sur les difficultés matérielles susceptibles d'entraver l'exercice effectif du droit de vote qui affectent les étudiants comme les jeunes travailleurs particulièrement mobiles. Enfin, au-delà des écoles, nous devrions aussi réfléchir aux outils à mettre en place pour renforcer la convergence des débats nationaux et européens dans nos assemblées comme dans les médias. C'est le sens des amendements que je défendrai pour modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui vise à renforcer les obligations des sociétés nationales de programme en matière d'actualité politique européenne. Lors des débats relatifs à la révision constitutionnelle, nous pourrons également proposer des solutions pour améliorer la coordination de nos travaux aux échelons national et européen. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, devant le niveau d'abstention aux élections européennes, chacun s'interroge sur la cause de ce fléau démocratique qui détourne les électeurs de leurs représentants. C'est la raison avancée, du moins par le Gouvernement, pour présenter le projet de loi que nous examinons. Il est vrai-chacun peut le mesurer-que la quasi-totalité des Français ignore qui sont leurs représentants au Parlement européen.

également, que les huit circonscriptions interrégionales actuelles n'ont guère de sens. Trop étendues, elles ne sont identifiées par personne, et surtout pas par les électeurs.

Il faut donc introduire plus de proximité. J'en viens à la solution retenue par le Gouvernement pour corriger cette situation : il propose de créer une circonscription encore plus grande, une circonscription unique. Puisqu'il y a un défaut de proximité, créons une circonscription encore plus étendue : telle est la solution paradoxale qui nous est soumise ! On aurait pu espérer un redécoupage des circonscriptions correspondant aux treize régions instaurées par la loi du 16 janvier 2015 C'est d'ailleurs l'objet de l'un des amendements que j'ai déposés, et qui vise à adapter le périmètre des circonscriptions régionales à la nouvelle carte des régions. Il faut toutefois relativiser l'amélioration de l'ancrage territorial que représenterait cette option compte tenu

faussement régionaux, nous aurons des députés européens encore plus irréels, en état d'apesanteur permanent faute du plus minime ancrage territorial. En fait, la création d'une circonscription unique aura bien une conséquence, mais celle-ci est déjà inscrite dans le mode de scrutin proportionnel : le renforcement naturel du poids des états-majors et des organisations politiques, au détriment des personnalités et de leurs qualités propres. En prétendant nationaliser les enjeux, vous ne ferez que placer les candidats sous le contrôle des partis et les candidats potentiels dans une situation de dépendance à leur égard.

que ce n'est là qu'une douce berceuse. Les exemples d'apparatchiks, de recasés et de recalés en tout genre abondent au Parlement européen et seront confortés demain.

Par conséquent, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'argument selon lequel le passage de la circonscription interrégionale à la circonscription nationale permettra de réduire l'abstention est une pure fantaisie. est une pure fantaisie. C'est illusoire ! En maintenant le mode de scrutin proportionnel, on ne fera qu'encourager les candidats sélectionnés à rester dans le moule des états-majors, à ne pas déplaire, à ne pas sortir de la ligne pour être sûrs d'être investis ou réinvestis le moment venu par leur parti dans une position éligible.

vous l'aurez compris, la vraie question est celle du scrutin proportionnel, qui rend possible cette situation de dépendance très forte au parti plutôt qu'aux électeurs et qui suscite forcément le désintérêt et l'abstinence électorale,

Je rappelle qu'il ne revient à chaque État membre de définir le mode d'élection de ses représentants au Parlement européen que de manière parfaitement théorique. L'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct donne en effet la possibilité à chaque État membre de constituer des circonscriptions, mais sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.

nous l'avons encore vu au mois de juin dernier : ce sont les électeurs qui choisissent ou qui éliminent les candidats. C'est le fondement du suffrage universel que de permettre un choix clair, sans que ce vote soit dénaturé par le filtre des organisations politiques.

et, sauf à croire à la chimie médicale, il relève de la poudre de perlimpinpin plutôt que du principe actif, capable de porter remède à un mal profond. Tout cela est moralement indéfendable, politiquement désastreux et désespérant pour l'enjeu européen.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi rétablit la circonscription unique comme cadre de l'élection des représentants de la France au Parlement européen, mais il est aussi marqué par deux atteintes atteintes fortes au pluralisme- j'y reviendrai. Lors des débats sur la loi du 11 avril 2003, qui instaura des circonscriptions interrégionales au nombre de nous avions vivement protesté contre une évolution que nous ressentions alors contraire aux intérêts de notre peuple et de notre pays. Selon nous, établir des circonscriptions interrégionales avait en effet pour conséquence de favoriser les plus grandes forces qui sont les seules capables d'assurer une présence européenne sur l'ensemble du territoire. Nous avions dit et répété avec quelques autres- trop rares -que les élections européennes ont pour objet la représentation de notre peuple au Parlement européen et non pas celle de telle ou telle région. Nous le savons bien, l'Europe des régions, à laquelle nous nous opposons, pour notre part, est de longue date la visée des partisans d'un fédéralisme absolu permettant, au nom d'une hypothétique souveraineté européenne, de briser les résistances nationales au projet libéral, qui- ne l'oublions jamais -fut gravé dans le marbre des traités européens année après année, malgré l'opposition exprimée de manière forte en 2005 en France et dans de nombreux pays européens comme l'Irlande, le Danemark ou les Pays-Bas. Deux autres raisons pourraient susciter un grand scepticisme à l'égard de la régionalisation du scrutin. La première est que l'on ne peut espérer faire du scrutin européen un enjeu national en le disséminant de la sorte, et la seconde, très importante, est que la très grande majorité des États membres de l'Union européenne avait fait le choix de la circonscription unique, ce qui est toujours

2014. Il est donc certain que la régionalisation n'a pas permis de remédier à une abstention massive. Quant à rapprocher les citoyens des élus, la bonne blague ! sont les électeurs qui connaissent, dans une région, les noms de leurs députés européens. Dans son discours sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron a dit sa volonté de revenir à la circonscription unique alors que, dans le même temps- comme dirait l'autre -, il ne dissimule pas, ou en tout cas masque très mal, sa vision purement fédéraliste axée en particulier sur la notion de souveraineté européenne. Il propose pourtant de revenir à une circonscription unique, qui,, permet de mieux exprimer la voix de la Nation. Or nous savons que La République En Marche n'arrive pas à s'implanter localement faute de militants et de structures. C'est une organisation totalement verticale, portée par le chef de l'État et les soutiens médiatiques. De ce fait, la circonscription unique sera donc utile pour Emmanuel Macron et les siens. On peut par conséquent légitimement se demander si la motivation électoraliste n'explique pas pour partie ce choix. choix. Il est également possible d'estimer que la pensée complexe d'un président conscient, comme il l'indiquait le 26 septembre dernier, de l'échec démocratique d'une avant-garde européenne imposant ses choix sans assise démocratique l'incite à utiliser le retour à la circonscription unique comme tremplin vers un dépassement fédéraliste des nations par le biais d'une généralisation des listes transnationales pour marcher vers une Europe politique. Comme je l'ai indiqué deux aspects du texte annulent, selon moi, l'avancée indéniable qu'aurait pu constituer le retour à la circonscription unique. En premier lieu, le maintien du seuil de 5 % pour accéder à la répartition des sièges.

que le seuil fixé pour accéder au remboursement des frais de campagne est de 3 %. Soyons cohérents : alignons ces deux chiffres pour favoriser le débat et la participation ! Le maintien du seuil de 5 % pour accéder à la est un élément décisif dans notre choix de rejeter le présent projet de loi, mais il n'est pas le seul. Ce texte substitue au temps d'égalité qui prévalait pour la campagne officielle des élections européennes le principe d'équité pour l'une des parts de la répartition, poursuivant en cela l'oeuvre déjà entamée lors du quinquennat précédent. Le dispositif proposé, complexe, favorise, d'une part, les partis dominants, et, d'autre part, l'influence des médias télévisés et instituts de sondage sur la vie politique. Le pluralisme et la démocratie sont gravement mis en cause par cette disposition, sentiment renforcé par l'ajout en cours de la discussion à l'Assemblée nationale d'un article- ou plutôt d'un cavalier législatif - instaurant le même dispositif pour les élections législatives. Pourquoi une telle précipitation ? Emmanuel Macron applique encore une fois son fameux « en même temps ». L'habillage paraît relever du bon sens démocratique, mais lorsque vous examinez le contenu, c'est un verrouillage sophistiqué du système que vous découvrez. Dans son discours à la Sorbonne,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 14 du traité fondateur de l'Union européenne dispose : « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union.

plus faible taux de participation, à une courte encablure derrière le score du scrutin de 2009 qui était le plus déserté de tous les scrutins européens depuis 1979. Les Français ne s'intéresseraient pas à l'Europe en raison du caractère trop lointain de ses institutions et de ses représentants. En 2008, les bons docteurs de l'époque pensaient avoir trouvé le remède : il suffisait de découper le malade en 8 grandes eurorégions, et le tour serait joué On allait ainsi rapprocher les eurodéputés de leurs électeurs, et ces derniers se rueraient de nouveau dans les isoloirs. Mais patatras, après trois scrutins sur le mode eurorégional, les chiffres sont sans appel : c'est non pas le malade qui était imaginaire, mais bien les médecins qui prétendaient le soigner. Ainsi, le taux moyen d'abstention lors des trois derniers scrutins européens est supérieur de plus de sept points à celui des trois précédentes élections qui se tenaient dans le cadre d'un collège unique. en cause n'expliquent pas tout, mais croire qu'on instaurerait de cette façon une plus forte proximité grâce à quelques eurodéputés dispersés sur de très vastes territoires a quand même de quoi faire sourire les sénateurs que nous sommes qui savent combien il est difficile d'être présent sur tout un département ! La réforme de 2003 était si judicieuse qu'elle a provoqué la dénationalisation du débat sur l'Europe. Les médias ont alors profité de la brèche pour réduire leur traitement des élections européennes, prétextant la démultiplication et l'extrême hétérogénéité des listes en présence. Sans un débat un tant soit peu médiatisé, il ne faut pas s'étonner de la faible mobilisation du corps électoral.

mais dans un pays où la loi impose la parité lors des élections et dans un scrutin où la proportionnelle est de mise, le décalage observé au final est pour le moins surprenant. L'explication tient encore un chiffre : 8, comme 8 eurocirconscriptions, ce redécoupage ayant accru la tentation des partis de placer trop systématiquement un homme en tête de liste à ces élections. Avec un, ou plutôt une circonscription unique au lieu de 8, les élections européennes de 2014 auraient conduit à élire plus de 48 % de femmes en France., le redécoupage en treize eurorégions métropolitaines, que certains ont proposé, aurait eu pour effet singulier de faire chuter la représentation féminine, sur la base des résultats de 2014, nettement en dessous des 40 %. Oui ! Le retour à une circonscription unique est plus juste et plus équitable dans le cadre d'une élection à la proportionnelle telle que décidée par l'Acte européen du 20 septembre 1976 dont les lois françaises du 30 juin et du 7 juillet 1977 ont transposé les dispositions Ce retour à la circonscription unique est aussi plus juste en matière de représentation des formations politiques ayant franchi le seuil des 5 % des suffrages exprimés. Car, de fait, la fragmentation en multiples eurocirconscriptions a pour effet mécanique de rehausser le seuil d'éligibilité des candidats, provoquant une sorte de prime majoritaire en faveur des listes réalisant les plus forts scores au détriment des autres. autres. Généralement en France, lorsqu'un gouvernement engage une réforme électorale, celle-ci n'est jamais dénuée d'arrière-pensées, et il est en fréquent que le parti au pouvoir fasse en sorte que le nouveau dispositif le favorise arithmétiquement. Eh bien, telle n'est pas la motivation de la majorité aujourd'hui ! En effet, le retour à la circonscription unique devrait procurer à La République En Marche et à ses alliés moins de sièges que ce qu'un découpage en huit eurorégions pourrait lui valoir, au regard des récentes projections électorales. Si nous proposons ce dispositif, c'est tout simplement qu'il est plus juste et plus équitable politiquement. Alors, à défaut d'avoir une arrière-pensée électoraliste, nous avons bel et bien une arrière-pensée politique : celle de remettre l'Europe- plus encore qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de l'an passé -au coeur du débat politique national. Bien évidemment, c'est risqué, mais nous n'avons pas l'intention d'esquiver ce défi majeur pour notre pays. Il n'y a que les batailles que l'on refuse de mener qui conduisent à coup sûr à la défaite. Ce que nous voulons, c'est plus et mieux d'Europe, en même temps que nous voulons plus de France en Europe ! Je conclurai mon propos en avançant un dernier chiffre : 24. En effet, 24 sur 27, c'est le nombre d'États membres qui procéderont aux prochaines élections européennes dans le cadre d'une circonscription unique si, mes chers collègues, nous adoptons ce texte. Avoir un mode de scrutin le plus harmonisé possible, c'était bien l'esprit qui présidait aux débats préalables à l'adoption de l'Acte européen de 1976. Nous avons là une belle occasion de parachever ce voeu. voeu. Ne nous en privons pas ! Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera résolument en faveur du présent texte. Mes chers

La séance est reprise.

Le sujet, triste litanie, est une fois de plus le massacre de nombreux civils syriens par une attaque aux armes chimiques dans la banlieue de Damas par les troupes de Bachar el-Assad. Triste litanie aussi que le déni des parrains russes du dictateur, complices et coupables, dont l'ambassadeur à l'ONU explique sans rire qu'il s'agit de, comme il l'a fait il y a quelques jours dans l'affaire du Novitchok à Londres. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a annoncé ce week-end que la France prendrait ses responsabilités pour faire respecter le droit international. Je n'interviens pas pour vous demander d'annoncer, monsieur le Premier ministre, que vous allez envoyer les avions et les bombes. D'abord, au cas où vous auriez décidé de le faire, vous n'allez évidemment pas prévenir. Par ailleurs, nous connaissons trop désormais les conséquences catastrophiques de certaines « guerres humanitaires » pour ne pas réfléchir à deux fois à la nature de notre réponse. Mais il faut se rendre à l'évidence : la même situation s'est présentée il y a un an. Les Américains ont alors frappé une base vide, un acte sans lendemain. Et les massacres ont recommencé ; et les gaz ont refait leur apparition. Ma question est la suivante, monsieur le Premier ministre y a-t-il un moyen pour la France et ses alliés de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces actes inhumains, et comment la France peut-elle agir face à un régime irresponsable soutenu par un membre du Conseil de sécurité ?

deux nouvelles attaques à l'arme chimique sont intervenues récemment. Avec ces deux attaques chimiques, c'est une nouvelle fois le droit international et l'expression de la plus simple humanité qui ont été bafoués. Ces atteintes sont dues au régime syrien et elles traduisent le fait que le régime syrien, le système auquel nous faisons face, faisons face, ne reculera devant aucune transgression pour obtenir ce qu'il cherche, c'est-à-dire la fin militaire de toute résistance ou de toute opposition.

Avoir recours à l'arme chimique, c'est fondamentalement transgresser l'ordre international ; c'est assumer une violation caractérisée du protocole de 1925, de la convention de 1993 et de plusieurs résolutions des Nations unies. Utiliser l'arme chimique, c'est dire quelque chose ; c'est faire quelque chose. Et je crains, monsieur le président, que notre réponse à l'utilisation de cette arme ne dise quelque chose sur nous, de notre réaction, de la capacité que nous avons et de l'engagement que nous avons à faire respecter un ordonnancement international fragile, c'est vrai, mais auquel nous sommes attachés. Face à ces événements qui, je veux le souligner, sont d'une extrême gravité, le Président de la République l'a dit, la France assume ses responsabilités. Nous avons saisi le Conseil de sécurité- il s'est réuni hier et se réunit de nouveau aujourd'hui -pour demander l'arrêt des hostilités, pour demander l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et pour insister sur la nécessité de créer ou, plus exactement, monsieur le président, de recréer un mécanisme d'enquête international sur les attaques chimiques. Pour ce faire, nous nous coordonnons évidemment étroitement avec nos alliés et nos partenaires, notamment les États-Unis d'Amérique. outre, nous agissons pour que jamais- j'y insiste : jamais -l'emploi d'armes chimiques ne puisse avoir lieu en se prévalant d'une impunité quelconque. est bien le sens de l'initiative qui a été lancée par Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en janvier dernier, pour faciliter l'identification des individus ou des entités qui collaborent à ces programmes d'armes chimiques. Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, je dirai que l'émotion et l'horreur que suscitent ces actes sont évidemment partagées sur toutes ces travées. Nous savons tous ici que la solution à la crise syrienne sera une solution politique : aucune autre solution ne peut durablement régler le problème syrien. syrien. Mais, monsieur le président, je veux le dire, il ne peut pas y avoir de diplomatie crédible si de telles atrocités ne donnent pas lieu à une réponse forte, à une réponse unie, à une réponse résolue de la communauté internationale.

que la France et tous les pays démocratiques parviennent par tous les moyens à rétablir le tabou sur les carnages causés par l'usage des armes chimiques. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, qui s'adresse à Mme Sophie Cluzel, concerne le quatrième plan Autisme, pour la période 2018-2022. Je tiens, tout d'abord, à souligner le montant budgétaire de ce nouveau plan, fixé à 344 millions d'euros, montant supérieur à ceux des précédents programmes. Toutefois, je suis aujourd'hui inquiet du décalage entre les annonces du Président de la République de faire de la prise en charge de l'autisme une priorité nationale et les moyens qui y sont consacrés. En effet, sur une durée de cinq ans, le montant alloué à ce nouveau plan est d'environ 69 millions d'euros annuels. Est-ce suffisant pour financer un programme ambitieux ? Un montant de 69 millions d'euros par an pour améliorer le diagnostic, alors que les centres de ressources autisme sont saturés et trop peu nombreux ?

69 millions d'euros par an pour proposer une offre médico-sociale et des services adaptés à plus de 600 000 personnes atteintes de troubles autistiques, alors que seulement un tiers d'entre elles disposent d'une prise en charge de qualité ? Et, je n'oublie pas la situation des 6 500 Français exilés en Belgique Mon énumération est loin d'être complète, mais vous comprenez bien que nos inquiétudes sont avérées. Madame la secrétaire d'État, pensez-vous que ce quatrième plan soit à la hauteur d'une priorité nationale ?

je sais votre engagement sur ce sujet et sur la politique du handicap en général. Au terme de neuf mois de concertation, la stratégie nationale pour l'autisme est à la hauteur des ambitions et des attentes des familles ; le Premier ministre l'a dévoilée vendredi dernier : on peut dire que cette cette ambition a été inégalée jusqu'à aujourd'hui, avec une augmentation de 60 % par rapport aux précédents plans. Nous ne parlons plus de plan ; nous parlons d'une véritable stratégie nationale, derrière laquelle, collectivement, le Gouvernement est engagé. Oui, nous allons mettre les moyens pour pouvoir intervenir précocement, surtout avec un reste à charge pour les familles fortement diminué : plus de 90 millions d'euros seront vraiment investis

depuis la maternelle, avec des équipes renforcées et des vrais parcours, jusqu'à l'université pour ceux qui peuvent y accéder. Oui, là aussi, c'est un investissement de l'enseignement supérieur pour pouvoir offrir aux autistes un vrai parcours de qualification, avec avec une recherche d'excellence, remise au coeur de notre politique publique : plus de 14 millions d'euros pour des cohortes d'excellence, des centres d'excellence, des profils de postes universitaires- plus de dix postes seront consacrés à la recherche non seulement fondamentale, mais aussi appliquée. Alors oui,

: la particularité des différents plans Autisme est que, souvent, nous n'avons pas les moyens de consommer les crédits. Le temps de la politique et de l'administration n'est pas le temps des familles.

Certes, mais ce débauchage nourrit l'inquiétude. Nous sommes nombreux au Sénat à nous préoccuper de la perméabilité de l'éducation nationale à l'influence des géants américains du numérique. Très bien ! Une série de contrats conclus avec Google et Microsoft sans même d'appels d'offres du temps de votre prédécesseur fait craindre une mainmise progressive de ces acteurs sur la vie de millions d'enfants et d'enseignants. Ne soyons pas naïfs ! Ces géants américains de l'internet mènent des stratégies d'influence avérées avérées et étudiées, parfois déguisées derrière le soutien à l'innovation pédagogique : Microsoft soutient le forum des enseignants innovants ; après la Grande École du numérique, voilà que Google va financer la chaire sur l'intelligence artificielle polytechnique. Est-il normal, par ailleurs, que des sorties de classe aient lieu dans des boutiques Apple ? Cela pose la question du respect de la neutralité du service public ! Au demeurant, vous en conviendrez, la place de ces écoliers serait plutôt au musée ou à la bibliothèque

La scandaleuse affaire Cambridge Analytica-Facebook vient démontrer que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'engagements, de promesses et de chartes, même si le règlement général sur la protection des données s'appliquera Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il est temps de clarifier la position de votre ministère sur cette question ? La parole

l'école, le collège et le lycée ne sauraient être considérés comme des lieux d'entrée et de sortie en la matière, avec la possibilité de puiser dans les données ; je serai extrêmement vigilant sur ce point. Il est possible que des situations de fragilité aient été causées dans le passé, mais je serai le premier gardien d'une solidité à l'avenir, avec le futur directeur du numérique. Les visites dont vous

Je vous remercie de cette réponse, monsieur le ministre. Plus largement, je veux souligner que, au moment même où Marc Zuckerberg est auditionné par le Congrès américain, il nous faut absolument renoncer à cette complaisance naïve que nous avons entretenue jusqu'à maintenant dans nos relations

Ces attaques ont causé un bilan encore provisoire, mais déjà terrifiant : au moins cinquante morts et un millier de blessés, des civils, des hommes, des femmes et des enfants. En 1925, en adoptant le protocole de Genève qui interdisait les gaz asphyxiants, la communauté internationale avait dit : « Plus jamais ça » En 1993, en adoptant la convention interdisant l'usage des armes chimiques, la communauté internationale avait encore dit : « plus jamais ça ».

ceux qui détiennent le savoir-faire pour développer ce type d'agents toxiques et ceux qui croient dans leur intérêt militaire de les utiliser. fait-il peu de doute que le régime syrien est derrière ces attaques. Qu'en est-il de la responsabilité des alliés du régime syrien ? On le sait aujourd'hui : pas un seul avion syrien ne décolle sans que les autorités russes Nous demandons donc à la Russie un comportement de responsabilité. C'est ce qui nous a conduits à saisir le Conseil de sécurité, lequel s'est réuni hier soir et se réunit de nouveau en ce moment. C'est ce qui conduit aussi le Président de la République à engager la concertation avec nos partenaires et nos alliés. Celui-ci s'est entretenu deux fois avec le président Trump et également avec la Première ministre britannique. La communauté internationale est aujourd'hui face à ses responsabilités. Nous devons ensemble, de manière unie et résolue, tenir nos engagements, tenir notre parole !

Les craintes que nous entendons souvent dans nos territoires ont malheureusement été corroborées par les propos de nos interlocuteurs. Il semble que nous allions vers des coupes budgétaires drastiques dans le budget 2021-2027 de la PAC. Le commissaire Günther Oettinger a ainsi publiquement évoqué la perspective d'une baisse de 5 à 10 % de ce budget, soit plus de 3 milliards d'euros de moins par an, un chiffre qui dépasse l'entendement. Qui plus est, s'y ajouterait, dans le cas de la France, l'impact des revendications des pays de l'est de l'Union européenne qui portent sur une harmonisation « complète et rapide » du montant des paiements directs. Dès lors qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle entre les États membres, notre pays ne peut qu'y perdre. Comment consentir de tels sacrifices lorsque 30 % de nos agriculteurs ont des revenus de l'ordre de 350 euros par mois ? Jusqu'à présent, le Gouvernement a toujours indiqué- je reprends les propos de la ministre des affaires européennes -que la France était prête à moderniser la PAC, mais pas à la sacrifier. Pour un groupe aussi attaché à la construction européenne que celui du RDSE, lequel a défendu sans relâche le bien-fondé d'une politique agricole commune ambitieuse, il n'est pas question de partager l'idée d'un quelconque renoncement en la matière.

je vous remercie de votre question, qui me permet de rappeler que la politique agricole commune est une priorité pour la France. Justement, nous nous rendons dans toute l'Europe pour porter et promouvoir la position française sur cette future politique agricole commune, que nous sommes en train de construire avec nos partenaires. Monsieur le sénateur, vous l'avez dit, nous souhaitons une PAC beaucoup plus ambitieuse, une PAC plus solide, une PAC qui préserve des filets de sécurité

Mme Esther Benbassa, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Ce matin, dans une tribune publiée par France Info, 425 enseignants dénoncent la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants et sa plateforme Parcoursup. Ils appellent au retrait de cette « réforme absurde » et expriment leur soutien aux étudiants mobilisés depuis des semaines.

Le diagnostic est pourtant simple : faute de places et de moyens, tous les étudiants ne peuvent être accueillis dans l'enseignement supérieur français. Quant au milliard d'euros évoqué par Mme la ministre de l'enseignement supérieur, destiné à la refonte du premier cycle, nul n'en a encore vu la couleur et aucun document budgétaire n'y fait référence.

pour les cheminots, les soignants, les avocats, les magistrats, pour tous ceux qui défendent le service public, allez-vous persévérer dans la stratégie du pourrissement et du clivage ou ferez-vous enfin le choix

Enfin, je voudrais rappeler que croire dans le débat, croire dans l'échange, croire dans la démocratie, c'est aussi entendre la voix du plus grand nombre, c'est-à-dire celle des étudiants qui s'expriment pour dire qu'ils souhaitent réviser et passer leurs examens. Ils veulent de la majorité des organisations syndicales des personnels et des étudiants qui ont approuvé la loi, et respecter le vote du Parlement, qui a choisi de supprimer le tirage au sort !

mille coups de fouet en place publique, pour ajouter à la souffrance physique de la torture, celle de l'humiliation. Il a été reconnu coupable d'avoir troublé par ses écrits « l'ordre public, les valeurs religieuses et la morale ». Cela en effet, les droits des femmes saoudiennes, la liberté de conscience et la liberté d'expression. Raif Badawi est même accusé d'avoir déclaré que les musulmans, les chrétiens, les juifs et les athées sont tous égaux. Bien entendu, il ne l'a jamais dit, sinon cela ferait de lui un apostat. Il a défendu un droit universel que revendiquent tous les défenseurs et militants des droits humains partout dans le monde : la liberté d'expression. Raif Badawi est devenu un symbole, celui de la liberté d'opinion dans des pays où règne l'arbitraire. Le prince Mohammed ben Salmane achève aujourd'hui sa visite officielle à Paris. J'ai cru comprendre que le Président de la République se rendrait prochainement en visite à Riyad. Monsieur le Premier ministre, au nom de Ensaf, sa femme, et de ses enfants qui vivent désormais au Canada, et au nom de tous ceux qui pensent que la France n'a pas que des contrats à vendre, mais qu'elle a aussi une autorité particulière à faire valoir en matière de droits humains, pourriez-vous nous dire si vous avez indiqué au prince Mohammed ben Salmane que la France et l'ONU considéraient que la détention de Raif Badawi était une atteinte aux droits fondamentaux et que sa libération contribuerait grandement à crédibiliser les faibles signaux que l'Arabie Saoudite nous envoie pour nous convaincre de ces évolutions

a été accusé d'apostasie et d'insulte à l'islam et a été condamné en appel à mille coups de fouet et à dix ans de prison Il est détenu dans l'attente du réexamen de son dossier par la Cour suprême saoudienne. Son avocat a également été condamné à une lourde peine. La situation de Raif Badawi a suscité une mobilisation internationale forte et légitime, animée en particulier par son épouse. Le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov en 2015.

Badawi est emblématique des obstacles que rencontrent au Moyen-Orient, et notamment en Arabie Saoudite, les défenseurs des libertés d'expression, de conviction et de croyance. Nous parlons de libertés qui sont fondamentales. Nous parlons de valeurs universelles. Cela est d'autant plus nécessaire au moment où l'Arabie Saoudite est engagée, sous l'impulsion du prince Mohammed ben Salmane, dans un ambitieux programme de réformes qui ne porte pas que sur l'économie, mais qui dit viser aussi à moderniser la société et à promouvoir un islam de tolérance et d'ouverture. C'est bien parti ! Ces questions et le cas de M. Badawi sont des sujets que notre relation avec l'Arabie Saoudite nous permet d'évoquer sans détour, et c'est ce que nous faisons ! La parole

Mme Anne Brugnera, députée de la quatrième circonscription du Rhône, organisait une réunion publique intitulée « Plan étudiant et réforme du bac, pour la réussite de tous et de chacun », en présence de son collègue député, M. Jean-Luc Fugit, et du chef du service académique d'information et d'orientation. Sur l'invitation apparaissaient les logos de l'Assemblée nationale, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et de l'académie de Lyon. La diffusion de cette invitation a été assurée par les lycées.

Mme le recteur l'a d'ailleurs confirmé la semaine dernière dans la presse locale. Outre la participation d'un fonctionnaire à une réunion dont le caractère politique est clair, ces deux éléments corroborent le fait que les services académiques assument la publicité d'une réunion politique. Permettez-moi encore une fois de m'étonner de ces méthodes d'un autre temps, dans une République qui se veut pourtant exemplaire ! Monsieur le ministre, ma question est simple : le principe de neutralité qui s'impose à nos services publics, et au service public de l'éducation nationale en particulier, existe-t-il encore ?

Il est tout à fait normal que des réunions soient organisées pour expliquer ce qu'il en est. Les parlementaires sont d'abord et avant tout- je pense que vous serez d'accord avec ce que j'affirme -les représentants de la Nation : toute réunion qu'ils organisent n'est pas forcément une réunion politique

Madame la ministre des outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont confrontées à une crise sans précédent, due à une pollution d'ampleur exceptionnelle liée aux algues sargasses en provenance du Brésil. Outre les effets désastreux de ces algues sur l'environnement et sur l'économie, c'est surtout à propos de la santé de nos concitoyens que l'inquiétude est grandissante. En pourrissant sur notre littoral, les sargasses dégagent du gaz d'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac.

la commune de Capesterre, située sur l'île de Marie-Galante, est vidée de son économie. Plusieurs hôtels ont fermé, les pertes sont inestimables. Dans cette crise qui dure depuis 2011, les départements français d'Amérique attendent de l'État un engagement tangible qui démontre que les mots « République » et « solidarité nationale » se conjuguent au présent en tout point de notre territoire. À ce jour, le ramassage des algues constitue le seul moyen d'action des autorités pour lutter contre ce fléau. La France doit peser de tout son poids sur la scène internationale pour faire appliquer le principe pollueur-payeur en remontant à la source de la pollution. Cette crise appelle la mobilisation urgente d'importants moyens de collecte des algues en mer, mais également d'information, voire d'évacuation des populations exposées. L'annonce récente d'une enveloppe de 500 000 euros pour les dépenses d'investissement et d'une somme équivalente pour les dépenses de fonctionnement paraît bien dérisoire lorsque l'on sait que, en 2017, une seule des six agglomérations que compte l'archipel guadeloupéen a mobilisé près de 700 000 euros pour accompagner les quatre communes qui la composent dans leur action de nettoyage des plages souillées. Malgré l'important engagement financier de la collectivité régionale auprès des communes touchées, l'ampleur du phénomène dépasse les seules capacités des collectivités.

plus régionale et nous devons travailler avec nos partenaires internationaux sur ces questions. Au total, vous l'avez dit, plus de 2 millions d'euros ont été mobilisés en Guadeloupe depuis 2015, par le ministère de la transition écologique et solidaire et par l'ADEME, sur ces différents projets. De son côté, le ministère des outre-mer a mis en place un fonds d'urgence de 1,5

en mars dernier, une réunion avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe aura lieu la semaine prochaine. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Monsieur le ministre, pour faire face à la grogne des collectivités locales, notamment des plus petites et des plus fragiles d'entre elles, avait indiqué devant les préfets, au mois de septembre dernier, que l'ensemble des dotations des collectivités locales seraient maintenues. « C'est un engagement pris, c'est donc un engagement tenu ; et il sera respecté », avait-il ajouté. Le pacte financier entre l'État et les territoires ne devait concerner que les 300 plus grosses collectivités représentant 80 % des dépenses locales. Les élus locaux avaient alors compris que l'État ne toucherait pas aux dotations des communes qui, jusqu'à présent, ont supporté l'essentiel de l'effort budgétaire. Le montant des dotations versées aux collectivités territoriales est désormais connu la DGF, est en baisse de 135 millions d'euros ; la répartition financière pénalise 22 000 communes, qui voient leur dotation forfaitaire diminuer de 5,8 % en moyenne.

En effet, face à cette crise d'austérité, de nombreux maires de petites communes nous ont déjà alertés sur la difficulté engendrée par cette nouvelle baisse de DGF. Cette dernière impactera durement les missions indispensables des petites municipalités. Comment pouvez-vous expliquer cette décision, monsieur le ministre ? Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de s'occuper vraiment du sort des communes qui, bien souvent, sont le dernier lien entre les populations et les pouvoirs publics ?

la part forfaitaire de la DGF fait l'objet d'un écrêtement destiné à financer d'autres augmentations de dotations, par exemple celles qui sont liées à une augmentation de population ou au renforcement de la péréquation.

La stabilité de la DGF au plan national est une réalité, madame la sénatrice. C'est le pacte financier du Gouvernement

Les propos présidentiels sur la nécessité de « réparer » le lien « abîmé » entre l'Église catholique et l'État constituent incontestablement une remise en cause de la loi de 1905, et il en aurait été de même pour toute autre religion. remise en cause particulièrement dangereuse dans un contexte où l'intégrisme religieux mine au quotidien le vivre ensemble dans trop de nos quartiers, où le communautarisme et la loi religieuse priment sur la loi républicaine, avec les conséquences désastreuses que chacun peut mesurer au jour le jour. Qu'il y ait chez l'homme une quête d'absolu, une recherche de sens n'est pas sujet à caution, mais ce n'est pas l'apanage des religions et bien des athées ont, heureusement, une vie spirituelle. Que, selon ses propos, « pour des raisons à la fois biographiques, personnelles et intellectuelles », M. Macron se fasse « une plus haute idée des catholiques » est son droit le plus absolu. Mais M. Macron est Président de la République française et sa fonction l'oblige, plus que tout autre, à ne pas amalgamer ce qui doit relever de la sphère privée et ce qui relève de la sphère publique. La question est donc simple, monsieur le ministre à quelle fin le Président de la République a-t-il délibérément franchi la ligne rouge ? Entend-il remettre en cause cette pierre angulaire de notre République qu'est la séparation des Églises et de l'État, ce qui constituerait un séisme lourd de conséquences, ou bien, plus prosaïquement, était-il dans des propos de diversion pour détourner l'attention médiatique des multiples crispations qui traversent actuellement notre pays ?

Mesdames, messieurs les sénateurs, la loi de 1905 avait initialement été portée comme une loi de combat contre les religions.

liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer la religion de son choix. Nous ne parlons c'est que la pratique de cette religion ne porte pas atteinte à l'ordre public. Il n'y a rien à ajouter ni rien à retirer à cela

La séance est reprise. Mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Irma Rapuzzi, qui fut sénateur des Bouches-du-Rhône de 1955 à 1989. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans le contexte troublé que nous vivons aujourd'hui en Europe, notamment après le Brexit, nous avons un besoin impératif de renforcer l'adhésion de nos concitoyens aux valeurs européennes, de mieux leur en faire comprendre les enjeux, sans en cacher, bien sûr, les défaillances. L'élection européenne est une occasion unique de débat, mais encore faut-il que nos compatriotes se sentent impliqués ... Le rétablissement de la circonscription nationale unique d'il y a quinze ans ne me semble pas la bonne réponse. Il affaiblirait la représentation des territoires dans leur diversité et renforcerait le poids des états-majors de partis politiques dans la sélection des candidats, au détriment des militants et des élus de terrain. Je me concentrerai, ayant peu de temps, sur un sujet spécifique : celui de la représentation des 2,5 millions de Français de l'étranger, prioritairement concernés par les enjeux débattus au Parlement européen, mais qui n'y ont jamais obtenu de représentation directe. En 1979, l'élection européenne avait été la toute première occasion pour eux d'exercer leur droit de vote dans un scrutin national. La représentation au Parlement européen est aujourd'hui la dernière frontière pour un exercice complet de la citoyenneté française à l'international, après que la révision constitutionnelle de 2008 a porté les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, après le Sénat. Leur représentation au Parlement européen, pourtant, devrait aller de soi. Les Français de l'étranger, qu'ils vivent sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors, sont les premiers témoins et les premiers artisans de la construction européenne. Le référendum dit de Maastricht avait suscité l'adhésion de plus 80 80 % d'entre eux. Leur expérience, leurs compétences seraient extrêmement utiles au débat européen et à notre pays. C'est d'ailleurs une revendication ancienne, portée d'abord par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, puis par l'Assemblée des Français de l'étranger. Dès 1997, Michel Barnier avait proposé la délimitation de vingt et une circonscriptions, dont l'une aurait représenté les Français de l'étranger. Pourtant en 2003, ces derniers avaient été privés du droit de vote à l'élection européenne. En 2009, nous avions demandé que les deux sièges d'eurodéputés supplémentaires attribués à la France, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, reviennent aux représentants des Français de l'étranger. J'avais même déposé une proposition de loi en ce sens en 2014. Il a finalement été décidé de rattacher arbitrairement les Français de l'étranger à la circonscription d'Île-de-France, sans leur donner de représentants spécifiques, et leur abstention a bien sûr été considérable. Aujourd'hui, le retour à une circonscription unique sonne le glas de l'espoir d'une représentation spécifique des expatriés au Parlement européen- sauf acceptation miraculeuse de l'un de nos amendements. Je ne peux que le regretter Le vote du Parlement européen du 7 février dernier confirme que les esprits ne sont pas prêts pour des listes transnationales, pourtant voulues, dès l'origine, par les pères fondateurs de l'Europe. Il faut bien sûr en tenir compte, mais soyons un peu ambitieux pourquoi ne pas introduire progressivement une toute petite dose de représentation transnationale, en réservant quelques sièges à des députés élus par des expatriés européens ? Cela consoliderait le principe de citoyenneté européenne et la possibilité de vote dans l'État de résidence. Auditionnée au lendemain de Maastricht, au nom d'une association de citoyens européens, par la commission des affaires institutionnelles du Parlement européen, j'avais déjà proposé cette circonscription spécifique transnationale à l'échelle européenne. L'idée avait été jugée enthousiasmante par la commission, qui trouvait que ce serait donner corps au principe de citoyenneté européenne, mais rien n'a avancé depuis ! Je rappelle que 13 millions d'Européens vivent dans un autre État que le leur, qu'ils sont très impliqués sur ces questions. Alors, bien sûr, le débat doit être conduit à l'échelle européenne, mais la France, qui a été pionnière de la représentation nationale de ses propres expatriés, s'honorerait, aujourd'hui, de promouvoir leur représentation à l'échelle européenne. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est ironique, au moment où le Gouvernement s'apprête à consacrer le principe de la différenciation territoriale dans la Constitution, que nous soyons réunis pour examiner un mode de scrutin non différencié Mais avant d'en aborder les conséquences, en particulier en outre-mer, je veux d'emblée affirmer l'appartenance de l'outre-mer à la République, tout en disant ma conviction que cette appartenance ne saurait avoir pour effet de gommer la réalité ultramarine. C'est pourquoi je plaide pour que la loi sécurise la représentation de chacun des trois bassins océaniques au Parlement européen, car il est, sinon hypocrite, du moins illusoire de renvoyer aux partis politiques le soin de désigner en position éligible des candidats ultramarins sur les listes. La notion de position éligible est juridiquement inexistante et politiquement approximative. Imposer une discrimination géographique parmi les candidats éligibles serait anticonstitutionnel. La seule garantie est donc celle de la loi. Le mode de scrutin actuellement en vigueur a deux vertus, que l'outre-mer partage avec la métropole. Sa dimension territorialisée favorise un lien- même ténu -avec l'Union européenne. Chaque scrutin européen étant l'occasion de déplorer le taux d'abstention, il est surprenant de revenir sur cette dose de proximité, alors que les institutions européennes souffrent tant de leur éloignement. Territorialiser le scrutin, c'est aussi être respectueux de l'expression de chaque territoire et, pour l'outre-mer en particulier, c'est faire écho à l'inscription et à la reconnaissance, au sein des traités européens, des statuts de région ultrapériphérique- article -et de pays et territoire d'outre-mer- articles 198 à 204 du même traité. Comment la France peut-elle demander à la Roumanie, à l'Autriche, à la Finlande ou à la Slovaquie de tenir compte de ses outre-mer, si elle n'en assure pas l'incarnation, avec des représentants ? Le Sénat sait d'ailleurs à quel point la vigilance s'impose. Par deux fois, sur l'initiative de la délégation sénatoriale aux outre-mer et avec le précieux concours de la commission des affaires européennes, il a dû alerter la Commission européenne par le biais de résolutions, l'une portant sur l'inadaptation des normes agricoles, l'autre lui demandant de tenir compte des outre-mer français dans les négociations d'accords commerciaux. L'Europe, largement source du droit aujourd'hui applicable, produit parfois des normes inadaptées aux contextes ultramarins, lorsqu'elles ne sont pas simplement inexistantes. Mais que ce soit par inadaptation ou par le silence des textes, c'est le développement même des outre-mer qui est entravé. C'est donc peu dire qu'il reste du chemin à parcourir et combien ce serait régresser de ne pas affirmer l'existence des outre-mer en leur garantissant une représentation. Au Parlement, la création de la délégation sénatoriale aux outre-mer a contribué à mieux faire connaître les problématiques ultramarines, mais il reste qu'il est encore largement procédé aux adaptations des textes à l'outre-mer au lieu de favoriser le débat parlementaire. Or la réalité commande de contextualiser toute politique impactant l'outre-mer, qu'elle soit nationale ou européenne. Pour ce faire, encore faut-il connaître le contexte ! Loin de moi, néanmoins, l'idée de penser que les Ultramarins ne se sentiraient représentés que par des Ultramarins. Il s'agit au contraire de ne pas prendre le risque de fragiliser davantage des territoires dont la situation nécessite une vigilance constante. Je terminerai, madame la ministre, en rappelant que, voilà moins d'une semaine, Mme la garde des sceaux, répondant dans cet hémicycle à une observation de notre collègue martiniquaise, a indiqué que la différenciation est une « exigence légitime » des collectivités ultramarines. Mes chers collègues, il vous sera donné ce soir l'occasion de mettre en accord les paroles et les actes Je vous remercie

lisibilité. L'élection majeure, dans notre pays, est l'élection présidentielle dont la circonscription est, par définition, nationale. Que nous

que les priorités soient fixées, que les moyens et ambitions soient définis dans un débat partagé par nos concitoyens.

et objectifs. En 2018, la souveraineté de la France trouve sa pleine expression dans la construction européenne.

vise à abaisser le seuil d'éligibilité de 5 % à 3 %. La fixation d'un seuil de représentativité est un correctif majoritaire à la représentation proportionnelle. Il peut être justifié d'un point de vue démocratique, dès lors qu'il s'agit de dégager une majorité de gouvernement ou de gestion. Toutefois, ce n'est pas le cas du Parlement européen, lequel reflète la diversité politique européenne et ne procède pas d'une logique de majorité gouvernementale. En conséquence, rien ne justifie d'appliquer aux élections européennes des règles conduisant à réduire le pluralisme de la représentation. C'est pourtant à cela que conduit un seuil de 5 %, comme l'a formellement reconnu la cour constitutionnelle allemande dans un arrêt du 26 février 2014. Jusqu'aux élections européennes de 2009, ce seuil de 5 % s'appliquait en Allemagne pour participer à la répartition des sièges. Dans une décision du 9 novembre 2011, la cour de Karlsruhe a jugé ce seuil contraire à la loi fondamentale, car méconnaissant les principes d'égalité des citoyens devant la loi électorale et d'égalité de traitement des partis politiques.

ne pouvait se justifier que si elle était nécessaire à la formation d'une majorité de gouvernement, ce qui, en l'occurrence, n'était pas le cas. Ce raisonnement s'appuie sur des principes démocratiques généraux dont on voit mal pourquoi ils ne s'appliqueraient pas au cas de la France. Dans ces conditions, le moins que puisse faire le législateur français,

cela a été dit, des milliers de nos concitoyennes et de nos concitoyens d'une juste représentation et appauvrit notre vie démocratique. Ce choix d'un seuil de 5 % place la France

En écartant de fait 15 % à 20 % des suffrages exprimés de la répartition, le système en place renforce le phénomène d'abstention déjà très fort en raison du rejet d'une Europe aux centres de décision éloignés, d'une Europe au dogmatisme libéral étroit qui maintient les pays européens sous le poids de l'austérité. Supprimer ce seuil serait une mesure de bon sens démocratique renforçant le pluralisme et le débat d'idées. À l'heure où la question démocratique se pose dans le cadre du débat institutionnel, le Sénat s'honorerait de voter cet amendement.

a souhaité limiter son intervention sur la loi de 1977 à la seule mise en oeuvre de la circonscription unique et aux conséquences qu'elle emporte, notamment- nous en reparlerons au cours de la discussion -sur les dispositions nouvelles répondant aux injonctions

Si nous sommes favorables à la circonscription unique, nous dénonçons que soit proposée en même temps la modification des règles de temps de parole lors de la campagne électorale, modification qui privilégie les seuls partis défendant une Europe fédérale. La circonscription nationale revenue et retenue pour les prochaines élections européennes, qui est le point majeur de ce texte, a pour mérite de rappeler que les élus au Parlement européen sont les représentants non de territoires ou de régions, mais bel et bien de la France et des Français, peuple un

Cette nationalisation du scrutin est un modèle retenu dans l'immense majorité des autres États membres. Nous sommes inspirés, pour une fois, de les rejoindre sur ce point. Cette nationalisation a aussi le mérite de clarifier les positionnements des grands partis nationaux qui « surfent » sur une ambiguïté et qui trompent les électeurs. J'en veux pour exemple nos chers collègues du groupe Les Républicains qui nous disent vouloir marcher sur leurs deux jambes, l'une libérale et l'autre conservatrice- entendre, sur les questions européennes : l'une fédérale et l'autre souverainiste. Mes chers collègues, sur un sujet aussi essentiel, ces deux jambes ne se complètent pas, ne se synchronisent pas : elles s'opposent et s'entrechoquent. Il vous faut donc choisir, à moins de manipuler, une fois encore, les électeurs. nous avons toujours été très clairs : nous sommes pour une Europe des nations libres et souveraines, une Europe au service des peuples et des nations. Contrairement aux fédéralistes, qui en appellent à une Europe de la trique, nous souhaitons une Europe qui cultive les relations bilatérales et multilatérales librement consenties entre les pays, des relations respectant libertés et souverainetés nationales. Malheureusement, ce texte est entaché d'une réforme du temps de parole durant la campagne qui n'est pas acceptable. Dès que la démocratie repousse, vous sortez, mes chers collègues, votre lame législative pour la faucher ! Cette volonté de transformer le temps de parole attribué de façon inégalitaire pose un vrai problème démocratique. Comble de l'ironie, vous proposez de répartir les temps de parole proportionnellement aux groupes politiques non de l'assemblée européenne, mais de l'Assemblée nationale. Encore un coup de Jarnac qui confirmera aux Français que votre Union européenne ressemble décidément à une Union soviétique européenne

le souhait de restaurer une circonscription unique pour l'élection de nos députés européens n'augure rien de bon. Ce choix, caressé par certains, n'est pas le mien. À une époque où l'on reproche aux élus de s'éloigner de leurs électeurs, je m'étonne que l'on prône une mesure qui conforte l'entre-soi. Je préfère des députés élus dans des circonscriptions, fussent-elles imparfaites, à des élus désignés dans une circonscription nationale, sans aucun lien avec leurs électeurs. À mes yeux, seul le Président de la République est légitime à être élu dans une circonscription aux dimensions de la France. Depuis 2004, l'élection des députés européens dans des circonscriptions a rapproché ces élus de leurs électeurs. Nos parlementaires européens ont bien « localisé » leurs actions. Les campagnes électorales européennes sont l'occasion de contacts des candidats avec leurs électeurs. Serait-il démocratique de revenir au ? Souhaitons-nous des meetings désincarnés, purement centrés sur les problématiques d'un parti ? Le militant que je suis n'a guère de sympathie pour ces campagnes, dont l'enjeu était de savoir si l'on figurait sur la liste ... La création de circonscriptions pour les élections européennes a été un progrès dans le rapprochement avec nos électeurs. Sous couvert de modernité, certains songent pourtant à revenir Enfin, à ceux qui affirment que les élus européens sont désignés par leur parti, on peut répondre que plus il y a d'enracinement, plus il y a de légitimité. Et plus il y a de légitimité, plus il y a de liens avec les électeurs. Un élu désigné dans un territoire, c'est aussi une garantie d'indépendance. Un élu dont la liste couvre la Nation entière sera dans une situation de faiblesse : il ne pourra guère s'appuyer sur les électeurs de son territoire ; il devra tout à son parti. Dans certains cas, il pourra même être dans les mains de l'exécutif. Il ne sera là que pour faire de la figuration. Il ne sera là que pour un sigle ou pour un logo, sans aucun lien avec son terroir. Son travail au Parlement européen ne fera l'objet d'aucun suivi. Je m'étonne que l'on tourne le dos, avec autant de cynisme, à ce qui permet à une démocratie de vivre. Dans le feuilleton de la rénovation des institutions, l'épisode proposé par le Gouvernement n'est pas l'avenir de la démocratie, mais le retour vers le passé. Pour ces raisons, je voterai contre cet article, conformément à l'intime conviction de mes collègues du groupe Les Républicains. La

l'adoption d'un mode de scrutin proportionnel dans une circonscription unique, l'engouement pour le scrutin proportionnel rejoignant d'ailleurs la culture de la gauche. Pourtant,

très satisfaisant. Nos députés européens ne sont pas assez identifiés, pas assez accessibles, ce qui contribue à creuser encore davantage la distance entre les citoyens et l'Union européenne.

! Si toutes les réalités du territoire et du peuple français ne sont pas portées par les voix françaises, alors le rejet de l'Union européenne sera beaucoup plus fort. Cela ne nous empêche nullement d'avoir un débat sur ce que doit être l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on est élu député dans une circonscription

présenté aujourd'hui constituerait un bouleversement, à la fois du découpage des circonscriptions électorales et de leurs modalités pratiques, concernant les prochaines élections européennes prévues en 2019. Outre l'article 1, qui conduit au remplacement des huit circonscriptions régionales actuelles, dont la circonscription de l'outre-mer, par une circonscription nationale unique, du texte prévoyait initialement que les circonscriptions nationales pourraient être remplacées par une circonscription européenne, avec des listes transnationales en fonction des dispositions prises par l'Union européenne. La circonscription d'outre-mer permet à nos territoires d'être représentés en bénéficiant de trois sièges. Sa suppression constituerait donc une bien mauvaise nouvelle, puisque les candidats ultramarins auront toutes les difficultés du monde à obtenir une place en position éligible sur une liste nationale ou transnationale. De même, il est à prévoir que les petits partis politiques seront écartés et devront renoncer à présenter des listes à cette élection, car les listes nationales ou transnationales favoriseront avant tout les grands partis, qui disposent déjà de moyens importants. C'est pourquoi mes autres collègues ultramarins socialistes et moi-même avons déposé des amendements

comme les grandes oubliées de la politique européenne. Les implications et les conséquences seraient catastrophiques pour la France et l'Europe, dans la mesure où nos territoires sont étendus sur près de 8 millions de kilomètres carrés dans trois océans. Ils cumulent à eux tous

madame la ministre, mes chers collègues, le présent article vise à revenir à la circonscription unique, qui était celle des scrutins européens de 1979 à 1999. Quand, en 2004, l'UMP et le PS ont mis en place huit circonscriptions, leur objectif était d'avoir des députés européens plus proches de leurs concitoyens, afin de lutter contre le désintérêt progressif et la méfiance exprimés par les Français envers par les Français envers l'Union européenne, tant par l'abstention que par la montée électorale des mouvements populistes et europhobes. Avec une abstention avoisinant les 54 % en 2014, et un Front national en tête, on peut légitimement estimer que cette stratégie a échoué. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec des circonscriptions sans aucune cohérence géographique, culturelle ni historique, mais aussi une Union européenne toujours plus lointaine et technocratique. Ainsi, voter le retour à une circonscription unique nous semble pertinent. Nous pourrions ainsi rendre plus claire et compréhensible la campagne électorale, tout en donnant une véritable dimension politique aux débats. Notre Union européenne, qui se meurt de son bureaucratisme et de son opacité, ne devrait en tirer que des bénéfices. Par ailleurs, ce scrutin permettrait le respect d'une proportionnelle intégrale, seul système à même de rendre possible la plus juste représentation

Nous souhaitons d'ailleurs que, à l'avenir, ce mode de scrutin puisse être élargi à toutes les échéances électorales, y compris nationales. Nous voterons donc contre l'amendement de suppression de l'article 1,

et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a réorganisé le territoire national en huit circonscriptions interrégionales, afin de rapprocher les élus européens de leurs électeurs et d'endiguer l'abstention aux élections européennes en favorisant

Cependant, le scrutin régional est la norme dans la quasi-totalité des pays européens de plus de 20 millions d'habitants. Il est au demeurant illusoire de considérer qu'un agrandissement de la circonscription permettra de susciter un surcroît d'intérêt de la part des Français pour les élections européennes. Le retour à une circonscription unique ne peut contribuer à renforcer le lien de représentation entre citoyens et élus au Parlement européen. Au contraire, ce choix aura pour effet d'affaiblir la nécessaire territorialisation du scrutin et, finalement, d'éloigner un peu plus les électeurs de leurs représentants.

Je le rappelle, 23 États sur 27 ont choisi une circonscription nationale unique. C'est une évidence, pour représenter la population d'un État,

11 rectifié. Par cet amendement, il s'agit de faire correspondre les circonscriptions électorales des représentants français au Parlement européen avec les régions administratives métropolitaines, auxquelles s'ajoute une circonscription ultramarine unique. Cette proposition a déjà été beaucoup critiquée. Pourtant, parmi les motifs ayant conduit, en 2015, à la création des grandes régions était souvent citée la nécessité d'accroître le poids en Europe des régions françaises. Dès lors, le scrutin européen doit être l'occasion d'achever le travail. Il faut ancrer les députés européens dans des régions gestionnaires des fonds européens et en charge d'une partie des problématiques de l'Union. Alors que, avec le découpage de 2004, les députés européens représentaient des circonscriptions multirégionales vides de sens, cet amendement vise à ancrer les députés européens dans des régions constituant un échelon administratif essentiel, celui des préfectures régionales, un échelon politique majeur, celui des conseils régionaux et, plus globalement, un échelon de plus en plus structurant dans l'organisation de la vie économique, sociale, culturelle et sportive du pays. Nos députés seraient donc en phase avec des régions ayant leurs caractéristiques et problématiques propres : régions de montagne, régions maritimes, régions à dominante agricole, régions en position de carrefour sur les axes de mobilité européenne, régions frontalières ou régions ultramarines. Ce lien est également le seul moyen de ne pas laisser en dehors de l'aventure européenne les territoires de la France périphérique, en dissolvant leur représentation dans des listes nationales. Choisir une telle option ne peut que contribuer à accentuer une fracture préoccupante avec la France des centres connectés à la dynamique européenne. Certes, de nombreux pays ont des circonscriptions nationales, mais ce sont pour l'essentiel des pays beaucoup plus petits que la France. Les pays européens les plus grands et les plus peuplés ont fait le choix, à l'exception de l'Espagne, d'un mode de scrutin régionalisé. Nous ne pouvons, mes chers collègues, risquer d'éloigner davantage nos concitoyens, en renonçant à toute incarnation territoriale. Un scrutin véritablement régionalisé est le seul moyen de sceller la nécessaire proximité entre les citoyens et ceux qui les représentent. L'Europe, comme la France, s'incarne dans les territoires.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale, les Français établis hors de France sont les tout premiers concernés par la construction européenne. Ils en vivent au quotidien les enjeux, en subissent les conséquences quand elles sont négatives,

Il est pourtant primordial qu'ils puissent continuer à défendre, à Strasbourg ou à Bruxelles, les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités. Créer une circonscription

Pour s'assurer que les trois océans - Atlantique, Indien et Pacifique - seront bien représentés, cet amendement prévoit la création de trois circonscriptions ultramarines, selon le périmètre des trois sections prévues à l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977.

ont également une forme d'outre-mer, celui-ci n'a pas la dimension ni l'importance des territoires ultramarins français.

que le message que nous portons en faveur de l'outre-mer peut trouver des limites constitutionnelles, au regard de l'égalité devant le vote.

qui est source de contraintes importantes, notamment lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles de droit parmi les plus progressistes du monde dans un environnement économique plus contrasté que celui de l'Union européenne. Il est donc nécessaire d'exercer une surveillance particulière lors de l'examen de textes européens susceptibles d'impacter plus durement ces territoires. Je pense notamment à la mise en oeuvre de la politique agricole commune, à la politique environnementale ou encore à la conclusion d'accords de libre-échange par l'Union européenne. Pour justifier son absorption par la circonscription unique, il a été argué que la circonscription d'outre-mer n'avait pas de cohérence dès lors qu'elle réunissait des territoires éparpillés dans l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique. Il est vrai que des différences existent d'un territoire à l'autre. Mais nous faisons face à des défis similaires ; c'est la raison pour laquelle les contours de cette circonscription n'ont, jusqu'à présent, pas été contestés par les populations concernées. Contrairement aux autres territoires de la République, seuls ceux de l'outre-mer sont soumis à un statut constitutionnel particulier. Cela devrait permettre de minimiser le risque d'inconstitutionnalité. d'inconstitutionnalité. Il s'agit ici non pas d'une revendication identitaire, mais de réalisme ! Comment s'assurer que l'Union européenne sauvegarde les intérêts des territoires situés à ses confins, même les plus éloignés, sans que ces derniers soient convenablement représentés ? Je regretterais que nous ne prenions pas la mesure du risque qu'une telle réforme représente pour ces territoires, dont la valeur stratégique pour la France comme pour l'Union européenne n'est pas encore suffisamment reconnue

transversale ». Elle est contradictoire avec le projet du Gouvernement. La commission s'est prononcée nettement en faveur de la circonscription nationale, donc contre le découpage en circonscriptions régionales.

qui touche au sens politique des élections européennes, si nous pensons qu'il y a une représentation de la France au sein du Parlement européen, tous les eurodéputés français représentent tous les territoires

Deuxièmement, il y aurait une différenciation forte, et sans doute trop forte du point de vue de l'égalité du suffrage, entre des régions auxquelles l'on reconnaîtrait une représentation spécifique-

du maintien d'une circonscription ultramarine. Nous avons effectivement constaté que cela emportait plusieurs risques juridiques susceptibles d'être sanctionnés par le Conseil constitutionnel.

l'autre régionale. Un décalage apparaîtrait ainsi entre la part, prépondérante, des députés européens élus dans la circonscription métropolitaine et les quelques représentants élus dans la circonscription ultramarine. ultramarine. Garantir la spécificité d'une représentation territoriale aux électeurs ultramarins, spécificité dont le reste des électeurs ne bénéficieraient pas, présente des risques en termes d'égalité des citoyens devant le suffrage. Et le découpage de la circonscription ultramarine en trois circonscriptions correspondant aux trois océans, Pacifique, Atlantique et Indien, présente des risques des risques majeurs d'inconstitutionnalité au regard des écarts substantiels de représentation qu'elle emporte. Ainsi, dans la section Pacifique, un député européen représenterait 570 000 habitants, contre plus d'un million dans les sections Indien et Atlantique.

Si le Conseil constitutionnel peut accepter de déroger au principe d'élections sur des bases essentiellement démographiques, il y a fort à craindre que tel ne serait pas le cas ici au vu, d'une part, des écarts ainsi créés et, d'autre part, de l'objectif du projet de loi : créer une circonscription unique, dans une telle hypothèse. Les écarts de représentativité entre les électeurs seraient accrus et susceptibles de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, toujours au regard du principe d'égalité. En outre, de telles circonscriptions ne laisseraient aucune place à l'opposition. En effet, en vertu du principe constitutionnel de répartition des sièges sur des bases essentiellement démographiques, elles ne compteraient qu'un seul siège. Les risques d'une censure sont dès lors accrus.

La création d'une circonscription ultramarine nuirait évidemment à l'intelligibilité du scrutin pour les électeurs. Elle créerait pour les populations d'outre-mer le sentiment

En outre, une étude comparée montre que d'autres États membres disposant de régions ultrapériphériques, certes peut-être pas aussi étendues, comme le

qui est représentée au Parlement européen. Et tous les territoires ultramarins font partie de la communauté nationale.

politiques et à ceux qui constituent des listes de faire en sorte de représenter aussi bien le territoire hexagonal que les territoires ultramarins. Je n'imagine pas

du 16 avril 2016. En vertu de cette dernière, le Sénat juge « indispensable que les élus d'assemblées ou de parlements des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d'outre-mer dotés de pouvoirs législatifs continuent à être représentés au sein du Parlement européen

nous serions aujourd'hui bien inspirés d'essayer de faire converger nos votes avec les dispositions de cette résolution, en particulier celles qui concernent la circonscription

le dispositif n'a pas été examiné par le Conseil constitutionnel et qu'il y aurait un risque de rupture d'égalité, voire de rupture du critère démographique. il s'agit d'une circonscription ; c'est la répartition des sièges qui se fait par bassin océanique. En matière d'intelligibilité, de loyauté, de clarté et de sincérité du scrutin, on ne fait pas mieux

m'exprimer sur la deuxième série d'amendements, pour une représentation équilibrée des citoyens européens que sont les Français habitant dans les territoires ultrapériphériques.

des atouts supplémentaires pour faire exister l'Union européenne dans les zones géographiques du Pacifique et de l'océan Indien, à proximité des grands continents et des lieux d'échanges internationaux, puisque tel est déjà le chemin, ou

La séance est reprise. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.

éloignement de l'Europe continentale, contraintes naturelles liées à leur insularité et à leur étroitesse territoriale, vulnérabilité climatique- cyclones, volcans, séismes -et écologique, ainsi qu'une dépendance économique à l'égard de quelques produits agricoles, tels que N'oublions pas également que certains territoires- Martinique, Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte -sont concernés par le POSEI dans le domaine de la pêche et de l'agriculture. Ce sont ces spécificités qui nécessitent la survie

Je pourrais adapter ce propos en disant que les meilleurs spécialistes des affaires ultramarines sont les Ultramarins eux-mêmes. Cette idée de double circonscription a été prétendument étudiée, puis écartée au motif que les populations d'outre-mer auraient le sentiment de bénéficier d'un traitement politique différencié auquel elles n'aspirent pas nécessairement et que les députés européens n'ont pas vocation à représenter un territoire en particulier, mais l'ensemble des citoyens. Madame la ministre, mes chers collègues, soyons sérieux ! Si le sujet n'était pas vital pour nos concitoyens et nos territoires, cet argumentaire prêterait à sourire. Nos populations méritent le respect, celui de leur pensée, de leur liberté de vote, de leur identité et de leur représentativité. Je vous le dis, ce projet de loi est l'annonce de désastres assurés. Les pays et territoires d'outre-mer sont associés à l'Union européenne. Ils ont accès, sous certaines conditions, au marché commun et bénéficient d'un soutien financier de cette dernière pour leur développement économique et social. Nos ressortissants possèdent la citoyenneté européenne et sont, à ce titre, électeurs et éligibles aux élections européennes.

si on n'a pas peur du suffrage universel et si on accepte de confronter les opinions des uns et des autres, il est évident qu'il faut mettre en place un scrutin proportionnel dans une grande circonscription. Car, alors, c'est la

qui veulent tronçonner le scrutin jouent en fait contre la Nation, contre l'idée française, contre la place de la France dans l'Union européenne. Moi, je ne suis pas partisan de dissoudre la Nation au profit de l'Europe. Or, tout le monde le sait, à un moment donné, les partisans d'une Europe fédérale ont joué la carte des régions contre celle des nations. Je suis

nous ne pouvons que déplorer. L'enjeu européen n'a rien à voir avec la région ; il y a d'autres instances pour celle-ci.

Bonhomme. Le Sénat ne peut pas tenir deux discours selon les scrutins. Nous sommes ici les défenseurs d'un lien de représentation entre les élus et les citoyens, lien que nous voulons non pas distendre mais resserrer. C'est la position que nous nous apprêtons à prendre pour les scrutins nationaux, qu'il s'agisse de l'élection des députés ou de celle des sénateurs. Nous

pour les élus nationaux du Parlement français ne serait-il soudain plus valable pour les élus français au Parlement européen ? C'est la même problématique ! Dans les deux cas, on peut soutenir que les enjeux ne sont pas locaux,

pour que nous soyons proches de nos électeurs, pour que nous les entendions et les écoutions, et pour qu'ils puissent nourrir notre réflexion.

de la situation juridique que nous avons à traiter ... Précédemment, on ne tenait plus compte de la Constitution ; maintenant, on ne tient plus compte des accords internationaux. Il y a un traité européen ! Vous ne pouvez pas changer le mode de scrutin sans l'accord de tous les pays.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

que celui déposé par mes collègues Brisson et Bonhomme sur la régionalisation du scrutin, mais il vise à dissocier les Français de l'étranger de la circonscription d'Île-de-France pour créer une quatorzième circonscription. Je pense que les Français de l'étranger regarderont tous très attentivement le résultat de ce scrutin. La

alors qu'ils peuvent déjà voter dans leur pays de résidence, me semble nier la citoyenneté européenne et l'engagement européen d'une très grande majorité des Français qui vivent hors de France.